Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je salue M. Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, présent en tribune. Le Le 23 juin 1894, le baron Pierre de Coubertin réunit à la Sorbonne les acteurs du sport mondial avec pour objectif de faire renaître les jeux Olympiques. En 1948, le Comité international olympique choisit de commémorer cet acte fondateur en organisant le 23 juin la Journée Olympique, qui est, depuis lors, célébrée chaque année. À cette occasion, et à un mois, jour pour jour, de l'ouverture des jeux de Tokyo, je veux apporter, au nom du Sénat, notre soutien aux 1 400 athlètes et accompagnateurs de la délégation française. Je veux adresser à l'équipe de France, à nos athlètes Olympiques et Paralympiques, un message d'encouragement, eux qui ont vu leur période de préparation aux Jeux perturbée par la crise que nous traversons. Le public français sera, comme lors de chaque olympiade, uni derrière ses champions, notamment au travers des nombreuses manifestations qui auront lieu sur l'ensemble du territoire. À l'issue de ces Jeux, le 8 août, la flamme passera de Tokyo à Paris pour la tenue, en 2024, du plus grand événement jamais organisé en France, qui est aussi une véritable chance pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, cela vous rappellera une mission que vous avez conduite Au-delà de nos athlètes, je veux adresser ici un message de sympathie à l'ensemble de la filière sportive, touchée par de longs mois de restrictions. J'ai à l'esprit notamment les associations, le sport amateur comme le sport professionnel. Tel est le message que je souhaitais vous adresser, mes chers collègues, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent sur Public Sénat, à l'ouverture de notre séance de questions d'actualité au Gouvernement. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, la commission des lois demande au Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, afin de mener une mission d'information sur les dysfonctionnements constatés dans l'organisation des élections départementales et régionales de juin 2021. La conférence des présidents a fixé à demain, dix heures trente, l'examen en séance publique de cette demande. Acte est donné de cette communication. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Chacun sera attentif

et Territoires. Cette question s'adressait initialement à Mme la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Ce week-end, un jeune rennais de 22 ans avait décidé d'aller danser. Après des mois de couvre-feu et de confinement, c'est à Redon, avec quelques centaines de jeunes, qu'il devait renouer avec la fête. Il y perdra une main, victime de la répression phénoménale de cette ; victime, une nouvelle fois, d'une grenade tirée de façon indéterminée dans la foule ; victime de méthodes de maintien de l'ordre placées sous le régime de l'escalade de la violence. En plus des atteintes aux personnes, les forces de l'ordre ont procédé à la destruction de 100 000 euros de matériel musical à coups de hache. Dans quel autre pays voit-on les forces de l'ordre détruire du matériel musical, avec autant d'acharnement, en dehors de toute procédure et s'en réjouir sur les réseaux sociaux ? L'absence de réaction du ministère de la culture démontre une nouvelle fois le mépris dans lequel celui-ci tient cette scène et la jeunesse. Il y a quelques semaines, lors de la présentation des protocoles sanitaires de déconfinement du monde de la culture, face à l'absence de perspectives pour les musiques actuelles et les concerts debout, je posais la question à Roselyne Bachelot : allons-nous passer un été culturel sous le signe de la répression ? Ce lundi 21 juin, premier jour de l'été, nous avons enfin eu la réponse plusieurs rassemblements festifs ont été dispersés sous des pluies de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Après un an et demi de confinement, la jeunesse de ce pays veut faire la fête, elle veut communier, mais n'a pas de perspectives claires. À l'Élysée, lundi, sous les dorures, on a pu danser avec Jean-Michel Jarre ; dans la rue, en revanche, on a matraqué et dispersé. Madame la ministre, ma question est la suivante : la politique culturelle pour la jeunesse est-elle sous-traitée à un ministre de l'intérieur, dont l'incompétence à organiser des élections n'a d'égale que son incompétence en matière de maintien de l'ordre ? Son approche répressive des rassemblements festifs, qui met en danger notre jeunesse, va-t-elle être revue ? Quelles sont les perspectives culturelles pour notre jeunesse cet été ? La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Monsieur le

le calme et l'organisation de l'intervention des forces de l'ordre. Certains individus ont d'ailleurs été secourus par des unités nautiques engagées dans ce dispositif, parce qu'il y avait, d'un côté, de l'eau, et, de l'autre,

et Territoires. Monsieur le ministre de l'intérieur, le spectre d'une abstention massive nous menaçait. Pour une fois, les sondages ne se sont pas trompés et l'ensemble de la classe politique a reçu une douche froide. L'abstention a atteint un niveau historique deux Français sur trois ne se sont pas exprimés. N'est-il pas urgent d'éclaircir les origines de ce phénomène et d'esquisser des pistes de réflexion, au-delà des satisfactions et des déceptions politiques des uns et des autres ? Le covid a sa part de responsabilité, certes, et le chemin vers les isoloirs n'était peut-être pas la priorité des Français. Si la grande gagnante est l'abstention, j'aimerais connaître la ou les sources de cet étrange paradoxe : il est très souvent reproché à notre classe politique nationale d'être éloignée du terrain ; mais quand vient le temps des élections locales, les électeurs sont aux abonnés absents. On a vu les « gilets jaunes » se plaindre du manque de représentativité ; on entend les jeunes se lamenter du manque de rendez-vous démocratiques, mais quand ces rendez-vous sont fixés, cela fait « pschitt ! », il n'y a plus personne pour les honorer. Comment expliquer cette désaffection démocratique ? Je n'ai pas d'explications satisfaisantes et les ratés de livraison des professions de foi ne justifient pas tout. Alors que nous disposons de moyens de communication vertigineux, je m'interroge sur les modalités de l'exercice démocratique. Aussi n'est-il pas temps de se poser officiellement certaines questions ? La concomitance de deux élections le même jour est-elle heureuse ? Ne serait-il pas opportun de recourir à des solutions technologiques face à un certain archaïsme démocratique, en admettant le vote par correspondance ou le vote par internet, même si beaucoup y sont réticents ? Ne faudrait-il pas se poser la question du vote obligatoire voire du vote blanc, même si cela ne s'inscrit pas forcément dans la démarche constitutionnelle ? Qui compose cette majorité silencieuse ? Après quarante ans de vie politique locale comme ancien maire d'une commune rurale et vingt années de vie parlementaire, je suis, comme nous tous, abasourdi

mais aussi par les politiques plus profondes qui touchent l'Occident, dans la mesure où tous les pays sont touchés, et singulièrement la France. Monsieur le sénateur, nous devons y réfléchir collectivement, après le second tour des élections régionales et départementales.

question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Des enveloppes de professions de foi dans les fossés et dans les poubelles, des enveloppes de professions de foi empilées sur les boîtes aux lettres des mairies, des enveloppes de professions de foi brûlées au coin des chemins, voilà la triste réalité d'une distribution chaotique et inadmissible des documents de propagande partout en France. Des millions d'électeurs n'ont reçu aucun des documents, pourtant indispensables pour les informer de la tenue des élections et pour éclairer leur choix. que la crise sanitaire a privé les candidats des moyens habituels de mener campagne, vous n'aviez aucun droit à l'erreur ! Dès lors que l'on fait du « quoi qu'il en coûte » son credo, on ne lésine pas sur les moyens. Après avoir affaibli le Parlement et ignoré les corps intermédiaires, après avoir favorisé le tirage au sort des concitoyens et l'établissement de conventions citoyennes, après avoir professé le « en même temps », qui contribue à donner le sentiment que, même si on élit quelqu'un, ce sont d'autres qui sont légitimes pour s'occuper de la

la vérité est que votre gouvernement est coupable. Coupable de ne pas avoir réagi en temps et en heure à un problème sur lequel vous étiez alertés depuis des semaines. Coupable d'avoir misé sur un coup de poker en choisissant une entreprise au bord de la faillite, pensant que l'abstention vous servirait, alors que celle-ci n'a finalement qu'amplifié votre élimination du second tour dans plusieurs régions. Coupable de jouer un jeu dangereux, en voulant réduire le débat démocratique à un affrontement entre saint Macron et le diable Le Pen. Alors que votre score aux régionales vous rappelle vos pires cauchemars, la droite républicaine, qui vous a mis au monde, n'est pas morte

tout à l'heure, nos collègues de la commission de la défense et des affaires étrangères, et son président, Christian Cambon, débattront avec vous, monsieur le Premier ministre, sur les conditions de la souveraineté française, sur sa remontée en puissance, sur la révision de la loi de programmation militaire et l'association du Parlement à celle-ci. Ils exprimeront probablement leur préoccupation quant à l'évolution des menaces et, en particulier, quant aux risques de conflits dits de haute intensité.

toutes ces questions sont interconnectées. Où en est, monsieur le ministre, la position française à l'égard de l'Iran ?

d'abord, les préoccupations que nous avons régulièrement exprimées à titre national, mais aussi avec nos partenaires européens, quant à la situation des droits de l'homme en Iran.

puisque les négociations sont engagées depuis plusieurs années sur la perspective d'un retour à la pleine mise en oeuvre de l'accord de Vienne sur le nucléaire.

La diplomatie française est donc pleinement mobilisée dans le cadre de ces négociations avec nos partenaires allemands et britanniques, ainsi qu'avec la Russie et la Chine et en lien étroit avec les États-Unis. Jean-Yves Le Drian rencontrera très prochainement à Paris son homologue américain, Antony Blinken, pour évoquer notamment la question des négociations sur le nucléaire. Nous souhaitons que celles-ci puissent aboutir rapidement, car le temps ne joue pour personne dans cette crise. Des décisions difficiles devront être prises dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines si elles ne devaient pas avancer. Au-delà de ces négociations sur le nucléaire, nous avons des discussions sur le retour des efforts de paix au Moyen-Orient, dans lesquelles la France est très impliquée. La parole

Pour le volet noir, pensons à nos concitoyens Fariba Adelkhah et Benjamin Brière, qui sont retenus dans des conditions insupportables. Pour le volet blanc, car il existe bel et bien, pensons au rôle décisif joué par les

pour tordre le bras des députés de votre majorité. Cette manoeuvre procédurale est d'autant plus scandaleuse qu'il s'agissait d'une journée réservée à l'initiative parlementaire et que la proposition de loi émanait du droit de pétition exercé par nos concitoyens. Sur le fond, vous avez surtout refusé de reconnaître l'autonomie des personnes en situation de handicap. En refusant d'individualiser le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), vous avez préféré renvoyer chaque personne dépendante du fait d'un handicap à une autre forme de dépendance, économique, vis-à-vis de sa compagne ou de son compagnon de vie. Cette humiliation pour la personne dépendante est pourtant dénoncée par l'ensemble des associations. Au nom de la responsabilité budgétaire, le Gouvernement s'enferme dans une posture bien éloignée des valeurs de progrès et d'humanité. Ma question est la suivante : allez-vous allez-vous inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire la proposition de loi qui reconnaît l'autonomie des personnes handicapées ou préférez-vous botter en touche en prétextant l'examen du budget pour voter un abattement fiscal

Non, monsieur le sénateur, notre approche n'est pas guidée par la seule volonté budgétaire. Elle est guidée par le fait d'assurer un système social fondé sur les principes de solidarité et de redistribution,

et plus de 180 euros de gain pour les couples dont le revenu du conjoint est situé autour du SMIC. Au nom des valeurs que porte votre groupe, vous devriez vous réjouir que l'on flèche l'argent vers ceux qui en ont le plus besoin et non vers les plus aisés, comme c'est le cas avec la déconjugalisation. Quand notre mesure ne fait aucun perdant, la vôtre prend l'AAH des personnes qui travaillent. Nous portons une mesure de simplification, une mesure de justice sociale. Je souhaite que le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale aboutisse. Parce que je crois à cette mesure redistributive qui est au coeur de notre ADN politique,

Le Président de la République a dévoilé, il y a un an, un plan de soutien inédit à la filière automobile, durement touchée par la crise, lequel prévoyait plus de 8 milliards d'euros d'aides, d'investissements et de prêts pour soutenir et accompagner la reconversion du secteur. C'est l'ambition du plan de relance : préparer la reprise en encourageant le développement de l'industrie de demain, tout en accompagnant celles et ceux qui font partie des secteurs sinistrés. Vendredi dernier, l'annonce du lancement du fonds d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile marque une nouvelle étape dans le déploiement du plan automobile. La signature de la convention entre les acteurs de la filière permettra de conforter le troisième volet du plan de soutien à l'automobile, annoncé au mois de mai dernier. Le ministre de l'économie l'a rappelé la semaine dernière à l'Assemblée nationale : avec le plan de relance, nous offrons une perspective aux Français, celle d'un redressement de l'économie en deux ans, qui doit nous permettre de retrouver en 2022 le niveau de développement économique de 2019, tout en accompagnant les emplois menacés vers les secteurs d'avenir. Madame la ministre, quelle est la place du fonds d'accompagnement dans cette perspective et comment pouvons-nous faire en sorte que les forces vives du secteur automobile soient au coeur de la reprise que nous appelons tous de nos voeux ?

Comme vous l'avez indiqué, face aux mutations de la filière automobile, nous devons tous nous mobiliser pour accompagner les salariés dans ces transitions. C'est tout l'objet du fonds d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile. Ce fonds, cofinancé à hauteur de 20 millions d'euros par les constructeurs Renault et Stellantis et à hauteur de 30 millions d'euros par l'État, permet de renforcer l'accompagnement des salariés des entreprises de la filière affectées par des restructurations. Il s'adresse particulièrement aux salariés des entreprises de la sous-traitance automobile en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces salariés seront accompagnés de manière renforcée par des cellules territoriales d'appui au reclassement. Concrètement, cela pourra se traduire par le financement de formations qualifiantes, par le versement d'aides à la création d'entreprise ou à la mobilité, ou encore par des primes au reclassement. Ce dispositif est d'ores et déjà mobilisé pour les salariés de MBF dans le Jura, dont je partage l'émotion à la suite de l'annonce de la liquidation de leur entreprise.

J'ai compris que vous faisiez référence à votre propre expérience, puisqu'en sus de vos fonctions de ministre vous étiez candidat deux fois aux élections de dimanche dernier Pendant ce temps, des élus de tous bords et de tous les territoires ont constaté que des plis non distribués avaient été jetés dans les fossés ou brûlés dans les bois. Le corps préfectoral lui-même nous a parfois fait part de sa honte au regard de l'image que l'État renvoie de lui-même. Vous répondiez dimanche en citant les chiffres communiqués par Adrexo, selon lesquels 21 000 plis n'auraient pas été distribués. Dans ma seule région de Bourgogne-Franche-Comté, j'aurais pu vous annoncer dès dimanche qu'on dépassait ces chiffres

; comme dans tous les bons questionnaires, plusieurs réponses sont possibles. Puisque c'est la faute de tout le monde, sauf la vôtre, monsieur le ministre, il reviendra à la commission d'enquête du Sénat de définir l'ampleur des dysfonctionnements observés dimanche. Dans cette attente, je vous poserai une question très politique de quel taux de non-distribution de la propagande électorale estimez-vous que votre propre responsabilité est engagée ?

Monsieur le ministre, votre responsabilité ne s'arrête pas à la question de la propagande officielle. Les sénateurs socialistes vous avaient alerté sur l'ampleur de l'abstention à venir. Nous avions proposé, dans cinq textes et au travers de trente amendements, des solutions alternatives, parmi lesquelles l'étalement du vote sur plusieurs jours ou le vote par correspondance.

dans les communes les plus rurales, les agences postales assurent les services de proximité, cette évolution est plus contestable dans des communes de 3 000 ou 4 000 habitants, sans oublier les fermetures surprises de certains bureaux, ou encore l'insuffisance de la compensation financière versée par La Poste aux communes pour les agences postales communales. En effet, selon le récent rapport d'information de nos collègues Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon,

227 millions pour l'aménagement du territoire et 260 millions pour l'accessibilité bancaire. Pourtant, monsieur le ministre, La Poste n'a reçu de l'État que 503 millions en compensation, ce qui représente un déficit de 1,6 milliard d'euros.

Malgré cela, La Poste connaît des difficultés. Le nombre d'objets, colis ou courriers qu'elle traite annuellement a été divisé par deux- il est passé de 18 milliards à 9 milliards entre 2008 et 2019 -et le nombre de courriers prioritaires adressés par les ménages chaque année a été divisé par Cela se traduit par des déficits et, partant, par la nécessité de réorganiser le service postal et de voir La Poste transformer ses métiers. Celle-ci s'y emploie, au travers d'une réorganisation territoriale, de partenariats accrus, mais aussi par la multiplication d'activités et par une forme de diversification.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là ? Nous avons atteint, dimanche, les taux de participation les plus bas de l'histoire de la République. À titre personnel, je n'ai pas à me plaindre, puisque, chez moi, nous avons remporté un large succès, fruit de notre travail au quotidien sur le terrain. Mais si l'on prend un peu de hauteur, il s'agit d'un vrai déni de démocratie, et vous avez, au Gouvernement, une lourde responsabilité. La première responsabilité est celle d'une campagne d'information minimaliste sur l'existence de deux scrutins locaux. Bien sûr, la réalité, c'est que vous êtes en campagne présidentielle. M. le Président étant en pleine tournée électorale, vous avez choisi de mettre ces deux scrutins d'ailleurs allés jusqu'à annoncer la date de la présidentielle entre les deux tours : c'est dire à quel point cela vous obsède ! Il est vrai que vous avez tout de même découvert le charme des Hauts-de-France :

Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. L'an dernier, les sinistres occasionnés par les intempéries ont coûté 1,5 milliard d'euros, un montant supérieur à la moyenne de ces quarante dernières années. Or la situation s'aggrave : je n'en veux pour preuve que les récentes inondations causées par de violents orages dans plusieurs départements, engendrant de graves dégâts et de nombreuses victimes. Les maires des communes concernées demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces conséquences croissantes du changement climatique mettent sous tension le régime dit CatNat et démontrent la nécessité d'assurer sa pérennité. À notre demande, une mission d'information

à mieux protéger et accompagner les victimes, à déplafonner le fonds Barnier et à renforcer le pouvoir des maires, toujours en première ligne dans ces circonstances. Malheureusement, ce texte n'a pas été soutenu par votre gouvernement, qui n'a pas souhaité l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le comble, c'est qu'un texte étrangement similaire a été déposé. Pis encore, le projet de loi Climat est totalement silencieux sur ces questions,

des sols est une des premières causes des catastrophes que nous vivons aujourd'hui. Je regrette d'ailleurs que, lors de l'examen de ce texte en commission, la territorialisation de l'objectif de division par deux d'ici à 2030 du rythme d'artificialisation ait été remise en cause par

En France, nous assistons à un rebond technique : après l'effondrement de 8 % du PIB, sa progression devrait atteindre 6 % cette année. Si une lecture partielle de la situation pourrait nous conduire à un excès d'optimisme, toute comparaison montre à quel point notre économie ressort de la crise plus dégradée que celles de nos voisins. Nos parts de marché à l'exportation régressent. « Ces chiffres sont mauvais », déclariez-vous en février dernier. En effet, pour l'année 2020, les chiffres publiés par la direction générale des douanes et droits indirects traduisent une inquiétante dégradation le déficit commercial de la France, qui était déjà de 57,9 milliards d'euros en 2019, atteint désormais 65,2 milliards d'euros. Les exportations françaises de biens et services se sont contractées plus fortement que dans les autres pays de la zone euro :-19,3 % pour notre pays, contre-13,2 % pour la zone euro. Le déficit commercial de la France s'est aggravé, pour atteindre 3,6 % du PIB, alors que les soldes de l'Espagne et de l'Italie s'amélioraient. Quant à l'Allemagne, elle maintient un excédent de 5,5 % de son PIB. La part de la France dans les exportations de la zone euro est à son plus bas niveau depuis vingt ans, et les chiffres de 2021 continuent à se dégrader. se dégrader. Plus grave encore, cette détérioration concerne la quasi-totalité des catégories de produits, y compris, désormais, le secteur agroalimentaire. Quelle conclusion tirer de ces résultats désastreux ? La compétitivité de nos entreprises s'est dégradée, la fiscalité française est plus que jamais désavantageuse par rapport aux autres pays, et notre industrie poursuit son érosion. Monsieur le ministre, le déclassement français est-il donc inéluctable ? Personne ne peut s'y résoudre. C'est pourquoi nous attendons des actions fortes de votre part !

La baisse de la fiscalité sur le capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production, le rapprochement des négociations au sein des entreprises du terrain, la simplification de la relation des entreprises avec l'administration, le paquet mis sur la formation professionnelle et sur l'innovation

Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques. Madame la ministre, depuis ma première mandature, soit depuis 2015, je suis continuellement interpellée par des fonctionnaires titulaires polynésiens qui émettent le voeu de rentrer servir dans leur territoire d'origine

certes intervenues, vous conviendrez qu'il est tout à fait normal, pour un enfant du pays, d'émettre le voeu de travailler dans la collectivité dont il est originaire, dès lors qu'il y a une vacance d'emploi correspondant à son grade dans son administration déconcentrée en Polynésie. Or force est de constater que, malgré la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

certains ministères techniques ignorent ce principe et privilégient l'affectation des fonctionnaires expatriés, au détriment de nos enfants ultramarins qui ont fait l'effort de passer les concours à l'échelon national puis de s'expatrier en métropole sans les avantages fournis uniquement dans le sens Paris-Papeete. De tels agissements de la bureaucratie parisienne nous laissent pantois en Polynésie et méritent d'être ouvertement dénoncés. Que comptez-vous faire, madame la ministre, pour que les fonctionnaires ultramarins soient définitivement considérés comme prioritaires quant à leurs voeux de mutation à destination de leur territoire d'origine ?

savez, depuis le début du quinquennat, le Gouvernement est entièrement mobilisé pour faire en sorte que la fonction publique soit plus représentative de l'ensemble des bassins de vie dont nous avons la responsabilité. C'est dans cet esprit que nous nous sommes engagés à faciliter, quand ils le souhaitent, le retour des fonctionnaires originaires des outre-mer dans leur territoire. Je tiens à rappeler un principe fondamental : comme tout fonctionnaire ultramarin pour son territoire, les fonctionnaires d'origine polynésienne sont bien prioritaires pour accéder aux emplois de la fonction publique en Polynésie. À cette fin, le critère du centre des intérêts matériels et moraux, le CIMM, que vous mentionnez, comme priorité légale d'affectation permettant le retour de nos fonctionnaires dans leur territoire d'origine, est particulièrement important. En tant que ministre de la fonction publique, je m'attache à promouvoir ce dispositif avec force auprès de nos agents publics. Comme le prévoit la loi de 2019, je vous remettrai, dans les tout prochains jours, un rapport sur ce sujet. sur ce sujet. Nous y dressons un bilan des dispositifs mis en place depuis 2017. Celui-ci montre que cette priorité légale récente constitue une véritable accélération des possibilités de mutation pour les agents qui les sollicitent. En effet, depuis 2017, les demandes effectuées au titre du centre des intérêts matériels et moraux aboutissent dans 28 % des cas à une affectation, soit un taux deux fois supérieur à celui des affectations attribuées au titre des autres priorités telles que la situation de handicap ou le rapprochement familial. Autrement dit, le centre des intérêts matériels et moraux est bien, dans l'application dans notre droit, la priorité des priorités. En Polynésie spécifiquement, il apparaît que certains agents qui souhaitent revenir ne recourent pas suffisamment à ce dispositif. Je m'attache donc, avec les employeurs publics, à faire en sorte que ces agents aient

En ayant recours au vote bloqué, vous avez empêché la tenue d'un débat légitime sur notre système de solidarité. Vous avez exprimé une nouvelle fois votre peu de considération à l'égard du Parlement, mais, surtout, à l'égard de tous ceux qui, depuis longtemps, se battent pour l'autonomie financière des personnes handicapées. En effet, le mécanisme actuel de calcul de l'AAH est injuste. Le bénéficiaire qui est en couple se voit privé de son allocation, dès lors que les revenus communs excèdent un plafond de ressources. Il se retrouve en situation d'extrême dépendance pour les dépenses quotidiennes. Je pense aux femmes handicapées, dont les revenus sont généralement plus faibles que ceux de leur conjoint. Je pense aux personnes qui font le choix de ne pas se mettre en couple pour ne pas perdre leur allocation. Je pense à ceux qui n'ont parfois d'autre choix que de se séparer pour retrouver leur indépendance financière. dernier, s'est prononcé en faveur de cette mesure de justice sociale, répondant au succès d'une initiative citoyenne sur la plateforme e-pétitions, voulue par le président Gérard Larcher pour établir un contact direct avec nos concitoyens. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre : allez-vous revenir sur votre position moralement regrettable, en acceptant enfin de supprimer les revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH ? La

je me demande bien ce qui a pu se produire entre le mois d'octobre 2018 et aujourd'hui, pour que votre groupe politique balaie d'un revers de main ses principes ... Permettez-moi de vous rappeler que, en 2018, dans ce même hémicycle, votre groupe affirmait, à propos de la déconjugalisation de l'AAH, la volonté de nier la situation familiale du bénéficiaire pour individualiser l'allocation participe de cette vision individualiste de l'homme et de la société qui tend vers un éclatement du lien social et une déconstruction de la famille ». Vous vous opposiez massivement, par principe, au nom des valeurs qui font la colonne vertébrale groupe, à la déconjugalisation de l'AAH et à ses effets. Vous vous refusiez à considérer la société comme une simple addition d'individus autonomes aux intérêts propres. Où sont donc passés ces principes de solidarité nationale et familiale, madame la sénatrice ? Considérez-vous à présent le couple comme une zone de violence permanente où les personnes en situation de handicap seraient systématiquement soumises ou sous emprise ? Parlons également de responsabilité budgétaire ! Vous vous érigez en permanence en garants du bon usage des deniers publics et vous passez votre temps à nous donner des leçons de gestion. Pourtant, vous êtes prêts à ouvrir la voie à la voie à un revenu universel sans condition de ressources et à élargir par conséquent ce principe au RSA, sur le budget des départements ! Pour rappel, le coût de la déconjugalisation du RSA est chiffré à 9 milliards d'euros. Si nous l'ajoutons à celui de la déconjugalisation de l'AAH, je serais très curieuse de connaître votre stratégie budgétaire.

Monsieur le Premier ministre, madame la ministre du travail, le 9 juin dernier, je vous interrogeais sur la réforme du chômage et ses effets dévastateurs pour les plus précaires. À cette occasion, le Gouvernement affirmait qu'aucun demandeur d'emploi ne serait pénalisé par cette réforme et qu'elle se justifiait par une situation économique favorable et un marché du travail en très nette reprise. Hier, le Conseil d'État a infirmé ces propos. Saisie par les syndicats, la juge des référés a suspendu le mode de calcul proposé par le Gouvernement et qui devait entrer en vigueur le 1 juillet prochain. La juge pointe les incertitudes économiques qui ne permettent pas la mise en place de ces nouvelles règles. Cette réforme rend moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés qui alternent contrats courts et inactivité. Ce nouveau contretemps pour votre réforme arrive après l'échec des négociations avec les partenaires sociaux en 2018. Malgré cet échec, vous aviez pris un décret, en juillet 2019, qui redéfinissait le régime d'assurance chômage.

Je rappelle que, d'après l'étude d'impact menée par l'Unédic, 1 150 000 personnes constateraient une baisse moyenne de 17 % de leur allocation, dont 345 000 jeunes qui peinent à trouver un emploi stable. Cette réforme est injuste et accentue les inégalités. Elle prévoit de faire des économies sur les chômeurs, en particulier sur les plus précaires. Nous vous le demandons à nouveau, monsieur le Premier ministre : abrogez une bonne fois pour toutes cette réforme injuste

aucun demandeur d'emploi ne verra son allocation baisser dans le cadre de la réforme. Le montant global des allocations est maintenu, et seuls les demandeurs d'emploi qui gagnent plus en étant au chômage qu'en travaillant pourront avoir, demain, une allocation plus basse, qu'au demeurant ils toucheront plus longtemps. Je vous invite à relire la décision du Conseil d'État. Elle ne remet absolument pas en cause la réforme de l'assurance chômage. ne retient aucun des arguments de fond soulevés par les organisations syndicales. Il nous dit que ce n'est pas le bon moment pour modifier le mode de calcul de l'allocation chômage, car, selon son analyse, la conjoncture économique serait trop incertaine. Pour ma part, je constate que l'économie repart et que les embauches sont très dynamiques. Je pense, madame la sénatrice, que vous entendez comme moi des chefs d'entreprise qui font état de difficultés de recrutement. C'est donc maintenant qu'il faut faire évoluer les comportements sur le marché du travail et qu'il faut lutter contre la précarité. De plus, je précise, puisque tout le monde ne semble pas l'avoir compris, que le bonus-malus entrera en vigueur dès le 1 juillet prochain pour les entreprises. Nous travaillons donc à rassurer davantage les acteurs, tant sur la situation économique que sur la dynamique de l'emploi. Nous préciserons, dans les prochains jours, les modalités d'une mise en oeuvre rapide de la réforme de l'assurance chômage. Dans l'immédiat, nous allons publier un décret pour prolonger les règles actuelles de calcul de l'allocation chômage, afin que les demandeurs d'emploi continuent d'être indemnisés après le 1 juillet. L'ambition du Gouvernement reste inchangée : accompagner la reprise de notre économie en répondant aux besoins de recrutement des entreprises et lutter contre la précarité, notamment grâce à une mise en oeuvre rapide de la réforme de l'assurance chômage.

Le plan de relance américain, une forte demande chinoise, et bientôt russe, dopent la demande de bois à l'échelle mondiale, avec pour effet une flambée des prix sans précédent, qui n'est pas sans conséquences pour notre pays. Des grumes et des sciages de chênes et de résineux sont trop massivement exportés, ce qui met en péril nos ressources nationales. Les prix s'envolent, car les traders étrangers ont des moyens financiers bien supérieurs à ceux des acheteurs français. Les professionnels de la construction bois, les charpentiers et les menuisiers de nos territoires ne peuvent plus honorer leurs commandes. Des chantiers se trouvent à l'arrêt, d'autres ne pourront démarrer comme prévu. Face à ce phénomène, il est essentiel de trouver rapidement des leviers d'action, même si nous savons que la situation est complexe et que les marges de manoeuvre sont limitées, eu égard à la réglementation européenne. La semaine dernière, dans le cadre des débats sur la loi Climat, un amendement visant à restaurer la carte professionnelle d'exploitant forestier a été adopté par le Sénat. Nous espérons que cette mesure sera maintenue lors des débats à l'Assemblée nationale.

des comptes publics. Madame la sénatrice Drexler, vous l'avez dit, la situation est complexe. Un certain nombre de règles, notamment communautaires, mais pas seulement, s'imposent à nous et encadrent la manière dont nous pouvons répondre aux problématiques de la filière bois.

à ne pas appliquer de pénalités sur les marchés qui seraient retardés par des problèmes d'approvisionnement. C'est ce que fera l'État, et nous avons invité les collectivités qui le souhaiteraient, dans le respect de la libre administration, à le faire aussi. Par ailleurs, nous sommes convaincus que la réponse ne doit pas seulement être conjoncturelle, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le cadre que vous avez évoqué. Elle doit aussi être de plus long terme, ce qui exige de développer des outils très transversaux.

Plus précisément, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe globale de 200 millions d'euros est consacrée à la création d'un Fonds forêt non seulement pour accompagner les propriétaires en matière de diversification et de renouvellement des parcelles, mais aussi pour accompagner la filière en matière de plantations et de graines, ou encore pour améliorer la connaissance cartographique de la forêt. Nous irons plus loin, puisque très prochainement deux appels à manifestation d'intérêt seront ouverts : le premier portera sur la construction bois carbone et le second sur le développement des produits bois et des systèmes de construction. L'objectif est de permettre à la filière bois française de s'adapter aux réglementations environnementales en matière de construction de bâtiments neufs et de renforcer cette chaîne de valeur de la filière forêt. C'est un travail de longue haleine. Les réponses conjoncturelles que j'ai évoquées

pour la réplique. En ce qui concerne la forêt publique, des mesures ont été prises pour garantir l'approvisionnement de la filière française, notamment par le biais de contrats d'approvisionnement ou de ventes labellisées de chênes. Cependant, plus de 60 % des stocks de bois privés français sont vendus à des professionnels pour être exportés. Il est capital Il est capital de trouver les outils qui permettront de réguler cet approvisionnement. La France doit peser de tout son poids au niveau européen pour que des mesures de préservation de nos ressources naturelles soient mises en place, afin d'échapper à la prédation de nos ressources forestières et à ses conséquences économiques et sociales, qui pourraient bien se révéler dramatiques. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour le groupe Union Centriste.

La construction des gendarmeries est assurée par des organismes dédiés comme Idéha ou Soderec, qui refacturent ensuite un loyer aux communes, loyer que l'État leur rembourse en contrepartie de la jouissance des locaux. Au début, l'opération est équilibrée, en grande partie, sinon totalement. Au fil du temps, néanmoins, ces deux loyers n'évoluent pas de la même manière. Le premier s'adosse à un indice BT01 du bâtiment, qui augmente, et le second à l'évaluation du service France Domaine, qui déprécie les immeubles et, donc, diminue les loyers de l'État au fil des années. En résumé, l'un monte quand l'autre descend. Très rapidement, une différence apparaît entre le loyer demandé par les organismes constructeurs et le loyer versé par l'État aux communes. Le manque à gagner constaté, par exemple, dans quatre communes du département du Doubs, Bavans, Bethoncourt, Étupes et Hérimoncourt, s'échelonne de 50 000 à 183 000 euros par an, ce qui représente pour l'une de ces communes une perte de plus de 1 million d'euros sur dix ans. Monsieur le ministre, avez-vous connaissance de cette situation ? Si oui, comment comptez-vous mettre fin à cet effet ciseaux préjudiciable aux finances des collectivités ? Pourquoi l'État ne payerait-il pas directement le loyer des gendarmeries aux promoteurs plutôt que de conserver la commune comme intermédiaire ? La parole

La séance est reprise.

L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote, en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative à la programmation militaire.

a traduit l'engagement pris par le Président de la République devant la Nation en 2017 de fixer une nouvelle ambition pour notre défense nationale et de restaurer les moyens qui lui sont affectés. Permettez-moi d'emblée de saluer, devant la Haute Assemblée, le travail de la ministre des armées, Mme Florence Parly, qui a élaboré, puis appliqué cette loi

Ce texte a fait l'objet d'un important travail avec le Parlement, tant lors de sa préparation que dans le suivi de son exécution. Je voudrais saluer tout particulièrement les sénateurs de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat qui y ont, notamment en 2017 et 2018, activement contribué. Le texte prévoyait que la LPM ferait l'objet d'une actualisation de façon à fixer, au-delà de 2023, la la trajectoire des ressources qui devaient permettre d'atteindre l'objectif fixé par le Président de la République, notamment celui de porter le budget des armées à 2 % du PIB à l'horizon de 2025. Il se trouve que la crise sanitaire, ou plus exactement ses conséquences économiques et financières, a significativement bouleversé le contexte dans lequel cette actualisation était prévue.

qui n'est, hélas ! pas complètement derrière nous -et ses conséquences économiques, dans un contexte qui reste incertain et que personne ne pouvait anticiper au moment de la préparation de la LPM, ont changé les conditions de cette actualisation et, donc, les perspectives pour 2024 et 2025, puisque tel est l'objet de ce

permettre à la France de retrouver un modèle d'armée complet et équilibré, à la hauteur des enjeux stratégiques d'aujourd'hui et de demain. Cette ambition est d'autant plus indispensable que nous sommes désormais confrontés à un « dérèglement du monde », pour reprendre les mots du chef de l'État. À la menace toujours présente du terrorisme, à cette menace qui relaie son obscurantisme par les réseaux de communication les plus modernes, tout en faisant appel à la technologie pour exploiter ou tenter d'exploiter les failles de nos systèmes de sécurité, à l'émiettement de la violence sans frein qu'elle provoque, s'est ajoutée la montée des appétits de certains pays en quête de puissance. Pour construire un modèle complet et équilibré, capable de faire face aux menaces d'aujourd'hui comme à celles de demain, le Président de la République a voulu donner l'impulsion nécessaire à une transformation profonde de nos armées. C'est ce qu'a traduit la loi de programmation militaire. Le premier objectif, le plus urgent, était d'abord de réparer les armées, dont les matériels étaient en mauvais état. La ténacité et le professionnalisme de nos soldats, marins et aviateurs, dont l'engagement est souvent allé bien au-delà de ce que prévoyaient

réparer pour rendre à nos armées les moyens de remplir durablement les missions qui sont les leurs. Le second objectif consistait à préparer l'avenir, c'est-à-dire à anticiper, moderniser et innover,

C'est avec la ferme volonté de réussir cette double opération de régénération et de modernisation que nous avons prévu une hausse historique du budget militaire. La force de nos armées et, donc, notre aptitude à rester maîtres de notre destin aux côtés de nos voisins européens et de nos alliés dépendent en effet de notre capacité à nous inscrire dans le temps long de l'histoire. À cet effet, il convenait d'abord de disposer de budgets en conformité avec nos besoins. Dans les dix années précédant le vote de la LPM en 2018, les crédits votés en loi de finances initiale dans le cadre de la mission « Défense » étaient quasi systématiquement inférieurs à ceux qui étaient prévus, cet écart pouvant aller jusqu'à 2,3 milliards d'euros pour une année donnée. Durant cette période, comme le Sénat l'a souvent relevé, ce ne sont pas moins de 3,8 milliards d'euros de crédits qui ont fait l'objet d'annulations ou de régulations pas moins de 60 000 postes qui ont été supprimés dans nos armées, si bien que notre effort de défense est progressivement passé de 2,1 % à 1,78 % du PIB en 2017. C'est à cette situation qu'il convenait de mettre fin ; ce que, ensemble, nous avons fait. Le budget annuel a en effet été porté, par la volonté de l'exécutif et par votre vote,

Très concrètement, après une augmentation de 1,8 milliard d'euros en 2018, ce sont des hausses de crédits de 1,7 milliard d'euros qui ont été confirmées chaque année. Au total,

soit plus de deux années de dépenses d'équipement, et une accélération sans précédent de l'investissement en faveur

dynamique, alors même que la crise sanitaire nous a par ailleurs conduits à puiser très significativement dans nos finances publiques. Je le dis, car certains pays se sont servis de leurs dépenses militaires comme variable d'ajustement. Tel ne fut pas le cas de la France. Aussi, je peux affirmer devant vous que les ressources et les objectifs de la programmation sont strictement respectés. C'est vrai ! C'est une réalité que vous me permettrez de qualifier d'historique, puisqu'il s'agit de la première LPM

Les premières mesures- vous y avez d'ailleurs contribué -ont été « à hauteur d'homme », selon l'expression consacrée. Elles ont permis d'agir sur le quotidien de celles et ceux qui choisissent le métier des armes. Ces mesures très concrètes visent en effet à améliorer leurs conditions de vie, d'entraînement et de combat. Ainsi, nous avons investi de manière inédite dans les infrastructures, notamment pour ce qui concerne le casernement.

Parallèlement, nous avons accéléré la modernisation des équipements. C'est notamment le cas de notre dissuasion nucléaire, dont le renouvellement des composantes aériennes et sous-marines est désormais engagé. Je fais aussi référence bien sûr aux nouveaux véhicules blindés conçus dans le cadre du programme Scorpion, qui renforcent considérablement la puissance de feu et la protection de notre armée de terre. Je pense encore à notre marine, à qui les nouveaux sous-marins de type Suffren, les Fremm- les frégates européennes multi-missions -, et, demain, le futur porte-avions vont permettre de faire face aux nouveaux défis posés par les perturbateurs de l'ordre international en mer. Je pense à notre armée de l'air dont la flotte d'avions de chasse et de drones armés se classera au meilleur rang mondial et qui a enfin pu renouveler son parc d'avions de transport et de ravitailleurs. Certains ont pu s'inquiéter ici même des retards qu'ils croyaient observer dans les livraisons de tel ou tel type d'équipement. Mme la ministre des armées pourra vous donner toutes les explications nécessaires, notamment les aléas qui en sont la cause. Ceux-ci sont d'une certaine façon la contrepartie d'une loi de programmation ambitieuse,

Ces variations sont finalement le reflet d'une gestion dynamique et réactive de la programmation. L'essentiel est que nos forces disposent des équipements dont elles ont besoin au bon moment, pour pouvoir s'engager Par ailleurs, et c'est un élément fondamental de notre politique de défense, la modernisation de nos forces doit s'accompagner d'une autonomie stratégique renforcée et d'un effort inédit en matière de renseignement. C'est évidemment dans ce secteur que la lutte contre le terrorisme exigeait un investissement majeur. Nous l'avons consenti : entre 2019 et 2023- permettez-moi d'anticiper le montant annuel moyen du budget consacré au renseignement sera d'environ 400 millions d'euros, contre 260 millions d'euros en moyenne sur la période 2014-2018. Nos services de renseignement verront leurs effectifs augmenter, puisque 25 % des créations de postes prévues par la LPM leur sont consacrées. De nouvelles capacités seront développées, en particulier pour intercepter les communications des groupes terroristes. le fonctionnement de nos services sera modernisé : la construction du nouveau siège de la DGSE, tout récemment confirmée par le Président de la République, en est une illustration emblématique.

L'accroissement du nombre de cybercombattants traduit notre volonté d'investir ce nouvel espace de conflictualité. Nous visons un objectif de plus de 4 000 au terme de la période couverte par la LPM. Le ministère dispose d'ores et déjà de 3 000 cybercombattants. Un pôle cyber des armées sera créé pour concentrer les expertises. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce nouvel élan donné à notre défense va évidemment de pair avec la volonté de la France d'amplifier la relance de l'Europe de la défense.

L'Union investit désormais directement dans les capacités militaires, ce qui constitue une avancée majeure dans sa prise en compte des enjeux de défense. Il en va de même de la Facilité européenne de paix, qui, soutenue par la France et approuvée par le Conseil européen le 22 mars dernier, a été dotée d'un budget à hauteur de 5 milliards d'euros : ce fonds témoigne de l'engagement collectif des pays de l'Union européenne à s'engager pour la paix et la stabilité internationales. Notre pays a donc joué un rôle moteur pour que des projets ambitieux soient lancés dans le cadre de la coopération structurée permanente, qui a donné lieu à la validation de quarante-six projets auxquels participent Avec nos partenaires européens, nous avons aussi lancé des programmes d'équipements stratégiques. Je pense en particulier au système de combat aérien du futur, qui associe la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ce programme ambitieux, qui combinera avions de chasse et drones d'accompagnement, donnera à nos pays et, plus largement, à l'Europe un avantage stratégique pour la maîtrise du ciel et les missions dans la troisième dimension. Dans le champ opérationnel, l'Initiative européenne d'intervention constitue un cadre souple pour réunir les nations qui veulent agir ensemble. Elle est en train de s'imposer comme une instance reconnue d'interopérabilité stratégique. Pour en revenir à la France, je veux insister devant vous sur les impacts de la loi de programmation militaire en termes de relance, d'industrie et d'emploi.

et 2022, qui correspondent à la période du plan de relance, ce sont 40 milliards d'euros qui seront investis dans nos entreprises et nos territoires, notamment à travers le plan de soutien aéronautique. Il faut ajouter à ces montants ceux qui sont liés à nos exportations d'armement, grâce auxquelles, entre 2018 et 2020, plus de 21 milliards d'euros de commandes ont contribué au dynamisme de nos régions. Comment ne pas insister devant vous sur les succès du Rafale à l'export, notamment avec les ventes récentes à la Grèce, à l'Égypte et à la Croatie, qui irriguent tout le tissu industriel de l'aéronautique de défense ?

par la direction générale de l'armement pour soutenir l'écosystème des industries de défense, si important pour notre souveraineté industrielle, avec une attention toute particulière portée aux petites et moyennes entreprises. Au total, les investissements prévus dans le cadre de la LPM vont contribuer à créer environ 25 000 emplois directs supplémentaires d'ici à 2022 et jusqu'à 70 000 à l'horizon de 2025. La seule industrie de défense représente près de 200 000 emplois de haut niveau, répartis dans toutes les régions- j'y insiste devant la chambre des territoires. rappelle également que notre armée est le premier service recruteur de l'État. Elle ouvre chaque année à des dizaines de milliers de jeunes le chemin de la compétence, de l'épanouissement et de la méritocratie républicaine. Enfin, comme vous le savez, elle reste implantée en de nombreux endroits de notre territoire national. Les objectifs visés par la loi de programmation militaire ont donc été pleinement respectés. Je tiens devant vous à saluer l'action, sous l'autorité de la ministre, du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et de la secrétaire générale pour l'administration du ministère des armées : ils ont tous joué un rôle décisif dans la mise en oeuvre de ce texte. Permettez-moi, dans cette circonstance réserver une mention spéciale au général François Lecointre, qui vit les moments ultimes de sa carrière militaire. L'évolution du contexte stratégique est venue confirmer la pertinence des priorités données à la loi de programmation militaire. Depuis 2018, la prolifération des armes nucléaires suscite à nouveau une inquiétude majeure. Les actes hostiles se sont multipliés dans les airs et sur les mers, par exemple en Méditerranée ou en mer de Chine. Certaines puissances régionales ont pris des positions stratégiques sans égard pour le droit international. Quant à la menace terroriste, je l'ai déjà évoquée, elle s'est diversifiée Les dispositions figurant dans la loi de programmation militaire doivent nous permettre de relever ces défis. Comme vous le savez, face à de nouvelles menaces, nous avons d'ores et déjà procédé à des inflexions, par à des inflexions, par exemple- je veux y insister devant le Sénat -en renforçant notre action dans le domaine spatial. La création d'un commandement interarmées dédié, l'effort que nous faisons pour pouvoir opérer dans l'espace, pour y surveiller nos adversaires, pour protéger nos satellites s'inscrivent dans cette projection déterminée vers un avenir qui ne peut se permettre de dupliquer ce qui existe déjà. Le budget d'équipement consacré à l'espace a ainsi été quasiment doublé depuis 2017. Les crises récentes et les leçons que notre pays a su en tirer ont conduit à des ajustements qui permettent désormais de détecter les menaces et de nous rendre plus résilients. C'est tout le sens des efforts que nous déployons pour accroître nos capacités opérationnelles, notamment dans les domaines prioritaires que sont le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique, mais aussi la santé, la lutte anti-drones et la lutte informationnelle. Nos forces, qui s'adaptent sans cesse aux menaces, sont fortement mobilisées, notamment pour lutter contre le terrorisme, tant dans le cadre d'opérations extérieures, au Sahel ou au Levant

Ne pas s'adapter en permanence au terrain comme aux circonstances revient évidemment à prendre un risque majeur. Cette règle, aussi ancienne que l'art de la guerre, est toujours d'actualité. C'est évidemment la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé la transformation de notre dispositif au Sahel.

force est tout à fait inédite : pour la première fois, des pays européens s'engagent ensemble, mais de manière autonome, dans des actions de combat. Nos partenaires et alliés ont ainsi compris à quel point la stabilité de cette région du monde

Cette évolution marque une étape significative dans notre engagement au Sahel. Le Gouvernement proposera au Parlement un débat spécifique sur le sujet. Je veux rendre hommage à nos soldats, marins et aviateurs engagés en opérations extérieures. Alors qu'une attaque au véhicule suicide vient de blesser six de nos soldats, en même temps que quatre civils maliens,

Nous leur en serons éternellement reconnaissants, car la France n'oublie jamais celles et ceux qui sont tombés pour défendre notre liberté et notre souveraineté. Mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à l'effort historique réalisé sous l'impulsion du Président de la République, nos armées ont pu être dotées de ressources à la hauteur de leurs missions et engager leur reconstruction et leur modernisation.

Cet effort, nous vous proposons de le poursuivre sans relâche ; de le poursuivre pour que notre pays puisse assurer sa défense et faire face aux défis qui viennent ; de le poursuivre, parce que sa longue histoire a appris à notre pays, de génération en génération, le caractère redoutable de ces défis.

C'est dans cet esprit que je me suis exprimé devant vous cet après-midi, un esprit d'union et de concorde, car, lorsqu'il s'agit de la souveraineté de notre pays et de la sécurité de nos concitoyens, lorsqu'il s'agit de la place de la de la place de la France dans le monde, je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités des sénatrices et des sénateurs. Aussi, la ministre et moi-même sommes particulièrement à l'écoute de vos contributions, analyses et propositions que ce débat permettra de mettre en exergue. À l'issue de ce débat, je vous demanderai par votre vote de renouveler l'engagement que nous avons pris en 2018 et de confirmer ainsi notre ambition collective, en matière tant de défense

à nos forces armées et à nos soldats grâce à cette loi de programmation militaire. C'est une question de sécurité, c'est une question de souveraineté, c'est une question qui fonde le rayonnement de la France dans le monde ! La parole

et inscrite dans la loi elle-même ne s'est pas franchement concrétisée devant le Parlement. Croyez bien que nous le déplorons. Est-ce parce que les circonstances ont changé ? Oui, les circonstances ont changé, mais dans un sens défavorable, avec la montée des menaces, la crise du covid-19 et la pression toujours plus forte sur nos finances publiques ! C'est précisément pour cela qu'il fallait une loi.

On ne trouvera pas plus de cohérence à cette décision en se référant aux orientations données par le Président de la République. J'ai assisté, à Brest, adressés aux forces armées ; je l'ai entendu saluer « le rôle essentiel de nos parlementaires qui, chaque année, veillent à la bonne exécution de la loi, protégeant nos propres engagements et notre capacité à affronter les défis de demain ».

Ce travail de six mois, que j'ai mené au nom de la commission, avec Jean-Marc Todeschini, a été réalisé grâce au soutien déterminé de nos huit rapporteurs budgétaires pour avis. Je veux ici solennellement les remercier, d'autant qu'ils ont travaillé dans des conditions difficiles, se heurtant souvent à un refus de communiquer un certain nombre d'informations. Or ce travail collectif a abouti à des conclusions importantes. Sur la forme, les enjeux de cette actualisation ne permettent pas, à l'évidence, de traiter cette dernière au cours d'un débat de deux heures, pas plus que lors d'auditions en commission. Sur le fond, la loi d'actualisation de la LPM, ce sont des chiffres et des tableaux, c'est la possibilité de creuser certains sujets, d'établir des priorités, d'identifier les retards, les redéploiements et les surcoûts et, donc, les économies à réaliser en fonction de ces priorités., c'est la possibilité d'amender le projet du Gouvernement projet du Gouvernement ... Je vous écoutais avec attention dresser ce bilan, certes élogieux, mais regardons l'avenir : vous ne proposez rien de tout cela, alors que c'est la norme démocratique dans tous les parlements et que vous l'aviez promis au Parlement, à nos armées et aux Français. Alors, de quoi parlons-nous ou, plutôt, de quoi aurions-nous dû parler ? Le Gouvernement a affirmé que la loi ne se justifiait pas, puisque, finalement, l'actualisation était modeste, portant sur 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la LPM. Pourtant, bien des éléments nouveaux sont survenus ces trois dernières années : l'irruption de nouvelles menaces, la cyberdéfense, l'espace, la nécessité d'accroître notre capacité en matière de renseignement, les retards des industriels, les conséquences de la vente des Rafale prélevés sur nos propres forces, le coût de la propulsion nucléaire du futur porte-avions de nouvelle génération, le coût des études, la commande non prévue d'une frégate de défense et d'intervention supplémentaire et, bien sûr, l'impact de la covid-19. C'est pourquoi, de notre point de vue, la réalité est tout autre : alors que nous n'en sommes même pas à la moitié de la LPM, nous avons chiffré le périmètre d'actualisation à 8,6 milliards d'euros. C'est huit fois plus que ce qui avait été annoncé

Ce n'était pas très aimable pour notre assemblée, mais passons ... Pourtant, nous avions fait le choix de retenir une estimation très prudente. Il faudrait y ajouter les chiffres que le ministère des armées ne nous a pas communiqués sur les sommes nécessaires, d'ici à 2025,

Quant à la régénération des véhicules blindés légers, notre commission ne cesse de vous alerter : ce sont 123 véhicules qui manqueront en 2025

Contrairement à ce que le Gouvernement a affirmé, la cible de 129 Rafale en 2025 ne sera pas atteinte : elle a été revue à 117 Rafale en raison du prélèvement des 12 appareils du contrat croate. Monsieur le Premier ministre,

Au-delà de ces grands programmes, d'autres sujets méritaient tout autant un examen attentif par le Parlement. C'est le cas du service de santé des armées ; voilà longtemps que nous alertons sur la centaine de médecins qui manque à ce service. Malheureusement, nos travaux ont révélé une aggravation de la situation situation : le déficit de 97 postes en 2020 est passé à 136 postes en 2021, en pleine crise du covid-19 ! Enfin, l'annonce de la fin de l'opération Barkhane, sans plus de précisions à ce jour, est évidemment un élément majeur de toute programmation militaire.

totalement ignoré cette disposition- nous le regrettons. Quelle sera la conséquence de la fin de l'opération Barkhane sur les crédits des armées ? Faut-il espérer un coût moindre ? Faut-il redouter à court terme un surcoût lié au démantèlement de certaines installations ? vous avez annoncé un débat ; il intervient bien tard, mais je le prends comme un signe d'espérance. En fait, on voit bien que, vu l'ampleur des sommes en jeu et la gravité des sujets, une loi d'actualisation était indispensable. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi y avez-vous renoncé ? Vous nous répondez : on ne connaît pas le PIB à l'horizon de 2025. Permettez-moi de vous le dire, c'est à la fois trompeur et inquiétant. C'est trompeur, car, le fond du sujet, ce n'est pas un pourcentage de PIB,

crédits est connu, nous l'avons discuté en 2018 : c'est une enveloppe globale de 295 milliards d'euros sur sept ans. C'est aussi inquiétant : en refusant de confirmer la trajectoire financière,

Monsieur le Premier ministre, les sénatrices et les sénateurs qui sont devant vous sont tous des élus de terrain. Nous savons bien quelle est la situation de nos finances publiques et de notre économie au sortir de la crise du covid-19. Oui, cet objectif de 295 milliards d'euros est difficile à tenir, mais il est indispensable : il y va de la sécurité des Français Or, pour que nos compatriotes acceptent de fournir cet effort, encore faut-il qu'ils aient conscience des enjeux et des choix à faire. Cette validation des choix ne peut prendre qu'une forme en démocratie : le vote de la loi par le Parlement.

mais écoutez bien ceci : le Sénat est une institution de la République dont la mission, quoi qu'il en coûte, est de contrôler l'action du Gouvernement. Sur la défense et les forces armées, le soutien du Sénat ne vous a jamais manqué. Alors, à votre tour, donnez-nous des preuves de votre respect pour le Sénat

pas d'armée, sans une solde ; pas de solde sans des impôts. » Tacite rappelait ainsi que la sécurité a un coût, auquel il est dangereux d'échapper. Après le démantèlement de l'Union soviétique, certains ont cru à un désarmement progressif, pensant qu'il suffirait d'engranger les dividendes de la paix en se plaçant sous le parapluie militaire américain. En France, nos armées ont trop souvent été la variable d'ajustement des politiques publiques. C'est ainsi que le budget de la défense est passé de 2,30 % du PIB en 2007 à 1,79 % en 2016. Or nos armées ont été constamment actives, tant sur la scène internationale qu'à l'intérieur de notre territoire. Nous voulons leur rendre hommage. Nos soldats, qui sacrifient jusqu'à leur vie pour la défense de la France, dont certains ont été récemment blessés au Mali, doivent avoir des moyens adaptés à leur mission. À cet égard, la loi de programmation militaire votée en 2018 marque un tournant que nous saluons à compter de cette date, la France s'est engagée à inverser la tendance et à renforcer ses capacités de défense. Cette remise à niveau s'appuie notamment sur une analyse exprimée dans la Revue stratégique, selon laquelle le monde dans lequel nous vivons devient plus instable et plus dangereux. La révision de cette analyse, au début de l'année, a été l'occasion de constater que les tendances envisagées en 2017 se confirment et qu'elles sont même en train de se réaliser plus vite que prévu. La France reste une cible privilégiée des djihadistes, en raison de ses valeurs et de son action en faveur de la liberté. Le retour des talibans en Afghanistan, accompagné par le retrait des troupes américaines, laisse craindre l'émergence d'un sanctuaire djihadiste. Au Sahel, territoire cinq fois plus étendu que l'Afghanistan, les islamistes gagnent du terrain. Notre armée doit également faire face à la menace grandissante exercée par des États qui emploient des stratégies hybrides à notre encontre. Ces derniers ont engagé un travail de sape de l'ordre mondial. Ils procèdent à des coups de force dès qu'ils le peuvent ; nous l'avons vu en Géorgie, en Ukraine, au Haut-Karabagh, en Méditerranée orientale, en Libye, au Venezuela ou encore en Syrie. Le plus souvent accomplies en zones grises, leurs actions franchissent parfois des lignes rouges : ce fut le cas avec l'emploi d'armes chimiques en Syrie, mais aussi lors d'assassinats au Royaume-Uni ou en Malaisie. La communauté internationale ainsi que les Occidentaux n'ont pas toujours su apporter les réponses adéquates à ces agressions. Et pour cause, les stratégies hybrides ont précisément pour objet d'être difficiles à attribuer et de se situer sous le seuil de déclenchement de riposte des pays ciblés. Ces États cherchent à affaiblir nos démocraties au moyen de stratégies indirectes ; ils manipulent l'information et tentent d'influencer nos élections. Nous devons nous donner les moyens de relever ce défi dans le cadre de l'actualisation de cette LPM. Ces agressions interviennent alors que les États-Unis ne consacrent plus autant d'attention à l'Europe. En effet, cela fait maintenant près de dix ans que le pivot américain vers l'Asie a été amorcé. Après une période de « mort cérébrale », le dernier sommet de l'OTAN a laissé espérer le retour des Américains auprès de leurs alliés. Il a surtout permis de confirmer que Pékin est la priorité numéro un de Washington. Dans cette perspective, il est indispensable que les Européens deviennent plus résilients. L'Union européenne est cependant encore loin de pouvoir assurer la défense de ses peuples. La France doit donc absolument adapter son modèle et se préparer à un conflit de haute intensité. En 2018, au-delà des clivages politiques, une très large majorité de sénateurs a soutenu l'adoption de la LPM. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de donner à nos soldats les moyens d'accomplir les missions qui leur sont confiées. Depuis 2019,

D'abord, parce que nous avons toujours eu à coeur de contribuer au mieux à la définition des efforts consentis par la Nation au profit de nos soldats, qui savent pouvoir compter sur notre entier soutien. Ensuite, parce que le parallélisme des formes imposerait que le Parlement actualise les lois de programmation qu'il a lui-même votées. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes félicité de la vente de Rafale à la Grèce, à l'Égypte et à la Croatie. Or le remplacement à neuf de ces avions représente un surcoût et un délai de livraison pour notre armée de l'air. L'incendie du sous-marin nucléaire d'attaque implique quant à lui un lourd prélèvement budgétaire. Le coût des OPEX, qui devait être pris en considération dans un cadre interministériel, et d'autres aspects cités par le président Christian Cambon conduisent à des dérapages budgétaires évidents nécessitant des arbitrages, qui méritent donc que le Parlement puisse jouer pleinement son rôle. La sécurité de nos soldats est prioritaire. Il ne faudrait pas que les petits équipements, notamment la rénovation des véhicules blindés légers, puissent être une variable d'ajustement. L'année 2020

Aucun parlementaire n'ignore que des choix délicats doivent être faits. L'existence de surcoûts et l'émergence de nouvelles priorités opérationnelles rendent les évolutions incontournables dans un contexte incertain. Vous l'avez rappelé, cette crise intervient à la fin du quinquennat. Le prochain Président de la République devra prendre des décisions dans un contexte que nous ne connaissons pas encore. Il devra notamment assurer la relance de l'économie, sans quoi rien n'est possible. Le chemin de crête est extrêmement étroit, car la relance ne doit pas oblitérer les autres priorités de notre pays, surtout en matière de défense. surtout en matière de défense. Or une grande partie des efforts de la LPM portent sur les dernières années de la programmation : 48 % du budget prévu par la loi de programmation militaire concerne le prochain quinquennat. Des arbitrages devront donc être décidés. Comme il s'agit d'arbitrages éminemment politiques, nous aurions souhaité que l'exécutif décide non pas seul, mais de concert avec la représentation nationale, comme ce fut le cas en 2015 pour la précédente LPM. À l'heure où le monde se réarme, tout retard peut mettre en danger la France et faire courir le risque de son déclassement. avez indiqué, monsieur le Premier ministre, plusieurs domaines prioritaires que nous approuvons : le renseignement, le cyberespace et le domaine spatial. Vous nous avez également invités à faire des propositions. propositions. À ce titre, je souhaiterais insister sur un sujet de première importance, alors que nous cumulons des retards. À l'échelle planétaire, la France est tenue d'exercer sa souveraineté sur 11 millions de kilomètres carrés d'océan. Les moyens que nous y consacrons sont-ils à la hauteur de ce défi ? Sommes-nous réellement en mesure de contrôler et de protéger nos intérêts ? Les Chinois et les Russes déploient des moyens considérables en mer. Or vous avez décidé de reporter d'un an le programme CHOF de renouvellement de la flotte hydrographique et océanographique. N'est-ce pas là un paradoxe ? Nous devrions au contraire accélérer la mise en oeuvre de ce programme. Je pense sincèrement que vous devriez revenir sur cette orientation. Il s'agit d'un enjeu majeur pour notre nation. Nous sommes en train d'accumuler un retard préoccupant au sujet des fonds marins. Le budget que nous consacrons à ce sujet est beaucoup trop faible eu égard à l'importance des enjeux. Vous ajoutez à la LPM une enveloppe de 40 millions d'euros, qui permettra de développer le prototype d'un robot sous-marin. Ainsi, nous commencerions à nous doter d'une capacité d'investigation à grande profondeur à la fin de

Dans cette vaste région du monde où les capacités militaires d'autres nations ne cessent de croître, un arbitrage à la baisse risque de nous être lourdement préjudiciable. En résumé, nous souhaitons que le ministère des armées soit conforté. Comme je le disais en introduction, notre sécurité a un prix ; la Nation, dans son entier, doit l'assumer. Tous les sénateurs de mon groupe soutiennent notre armée et les objectifs de la LPM. Néanmoins, certains s'abstiendront en raison de l'absence d'actualisation par une loi. La

Il y a trois ans, lors de l'adaptation de la loi de programmation militaire pour 2019-2025, le groupe écologiste n'existait pas au Sénat ; il n'a donc pas pu se prononcer sur les orientations de ce texte. donne l'occasion de nous exprimer : nous la saisissons volontiers, non sans amertume, car nous constatons qu'à rebours des engagements pris en 2018 par le Gouvernement, inscrits noir sur blanc à l'article 7 de cette loi, ce débat n'est, hélas ! qu'un ersatz du véritable contrôle parlementaire que nous devrions exercer. exercer. Sur ce point, je ne m'étendrai pas trop, mes chers collègues, car si nos visions de l'appareil militaire divergent, nous partageons aujourd'hui cette amertume, cette incompréhension, voire cette colère face aux manquements du Gouvernement. En effet, lorsque ce dernier a présenté il y a trois ans une programmation militaire très ambitieuse- j'y reviendrai -, le Parlement a fait le choix de soutenir cet effort budgétaire exceptionnel, sous la condition d'un contrôle renforcé et d'une exigence de transparence, et ce notamment en cas d'adaptation de la LMP au contexte sécuritaire et économique. Depuis 2018, l'évolution du contexte international n'a rien eu d'un long fleuve tranquille. Nous avons connu une pandémie, une crise économique mondiale, des changements majeurs dans notre engagement au Sahel, l'accélération des développements technologiques, la réapparition de conflits armés ouverts dans le Caucase et au Proche-Orient et l'accroissement des tensions à l'échelle mondiale. Comment croire que de tels bouleversements n'affectent pas profondément nos orientations stratégiques ? En toute cohérence avec les évolutions du contexte international, les ajustements de la programmation militaire sont nombreux. Dès lors, pourquoi insister sur la mise en oeuvre « à l'euro près » de cette programmation, selon les éléments de langage ministériels ? Nous savons pourtant, grâce à un travail important de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, que je tiens à saluer, que cette trajectoire budgétaire n'est respectée qu'en apparence. Ainsi, les calculs de la commission permettent d'affirmer que le périmètre budgétaire d'actualisation, qui aurait dû faire l'objet d'un examen parlementaire, serait non pas de 1 milliard d'euros, comme annoncé, mais de 8,6 milliards d'euros. Sur cette enveloppe considérable, le Parlement, hélas ! ne se prononcera pas. Cette mise à l'écart est inacceptable. De surcroît, nous sommes très inquiets des arbitrages qui seront faits ou qui ont déjà été décidés. Le renforcement de l'effort en faveur de certains programmes indispensables- spatial et programme numérique -ou plus discutables- propulsion nucléaire du futur porte-avions et cession de Rafale à la Croatie et la Grèce -pénalise d'autres programmes pourtant prioritaires, affectés par des économies et des reports. Dans un premier temps, nous alertons le Gouvernement sur la fragilisation des programmes qui touchent directement les conditions de vie et de travail du personnel de nos armées, programmes qui avaient permis de dire de cette LPM qu'elle était « à hauteur d'homme ». Certes, nous saluons Certes, nous saluons l'ajustement de 240 millions d'euros fait en faveur du plan Famille en 2019 et en 2020, mais, en parallèle, un nombre important de programmes qui touchent directement la protection, la sécurité et le bien-être de nos soldats, notamment ceux qui sont engagés en OPEX, ont fait l'objet de renoncements. J'en veux pour preuve l'abandon de 123 véhicules blindés légers par rapport à l'objectif initial. Du fait de leur mission de reconnaissance et de liaison en OPEX, ces véhicules sont très exposés aux mines et aux engins explosifs improvisés. Leur rénovation est donc essentielle pour la protection de nos soldats. Les objectifs relatifs au parc de véhicules blindés multi-rôles, comme le Griffon- eux aussi assurent la sécurité des soldats en OPEX -, déplorent également le manque D'autres aspects de la vie de nos forces armées, et pas des moindres, restent encore délaissés. L'effort en faveur du service de santé des armées semble trop faible alors que les départs de médecins des forces, dus notamment au manque de moyens et à la sursollicitation, sont nombreux.

Pour ces personnels, comme pour l'ensemble du corps médical des forces armées, on se demande encore par quels moyens le ministère entend lutter contre le. En 2020, le rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire confirmait que le nombre de départs dans les forces armées restait particulièrement élevé. sont pas épargnés ; ils quittent les armées notamment en raison de logements inadaptés à leurs besoins, ou simplement défaillants. Le groupe écologiste soutient donc des efforts plus importants en faveur des infrastructures, des équipements et des services essentiels aux conditions de vie et de travail de nos forces armées, ainsi que du personnel de santé. En second lieu, nous formons le voeu que les programmes faisant l'objet d'une coopération européenne, comme le système de lutte anti-mines du futur (Slamf), ne soient pas sujets à des reports, à l'heure où la construction de l'Europe de la défense est un enjeu crucial.

en particulier quand le spectre opérationnel s'élargit à de nouveaux espaces de conflictualité comme le numérique ou le spatial- vous l'avez rappelé, monsieur le Premier ministre. Dans l'équilibre actuel des grandes puissances mondiales, nous devons penser à l'échelle continentale. Une coopération systématique entre les armées européennes permettrait à la France, en allant au bout du pari de l'interdépendance communautaire européenne, de dépasser l'idée selon laquelle nous pourrions prolonger indéfiniment ce coûteux modèle. C'est précisément ce que nous enseignent les ajustements dont nous débattons : le déploiement accéléré de programmes à effet majeur dans ces nouveaux espaces de conflits se répercute sur les investissements nécessaires à l'entretien et à la modernisation du reste de notre appareil militaire et sur l'attractivité des métiers de nos armées. C'est donc en partie pour des raisons financières que la France doit se projeter davantage dans une stratégie pleinement continentale, en recherchant activement des coopérations européennes pour l'ensemble de ses programmes. de cette question financière, l'Europe de la défense est essentielle dans le contexte actuel de reconfiguration de l'espace mondial. Cette Europe de la défense doit aller au-delà du seul financement du développement de technologies et de capacités militaires.

alors que nous nous engageons dans un renforcement de notre système de dissuasion nucléaire. Ne devrions-nous pas, à l'inverse, engager une discussion commune afin de progresser vers la réduction de nos arsenaux respectifs, dans l'esprit du traité sur la non-prolifération des armes

Au milieu du gué, il nous paraît de toute façon difficile de revoir à la baisse la trajectoire budgétaire prévue : il ne faudrait pas reculer encore au détriment de programmes essentiels déjà pénalisés par vos arbitrages. par vos arbitrages. Voilà esquissée notre contribution au contrôle parlementaire qui aurait dû avoir lieu. Le Gouvernement ayant décidé de s'affranchir de la loi malgré les innombrables éléments qui nécessitent une actualisation législative, nous voterons contre cette déclaration.

Du Proche-Orient au Sahel, où nos troupes continuent de se battre, le changement climatique et son cortège de sécheresses et de catastrophes naturelles sont et seront à l'origine de l'immense majorité des conflits armés. Cela vous paraîtra peut-être encore suffisamment éloigné de vos propres vies pour que vous ne vous en alarmiez pas outre mesure. Mais, mes chers collègues, peut-être avez-vous lu vous aussi le document du Groupe d'experts Peut-être avez-vous lu ces mots : « Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants bien plus que sur la nôtre. » Dès lors, peut-être entendrez-vous notre appel : nous ne pouvons miser sur la montée en puissance de notre seul appareil militaire pour assurer la stabilité de la France et de l'Europe dans les prochaines décennies.

dont les montants paraissent bien dérisoires par rapport aux dépenses de défense. Pourtant, en luttant contre la raréfaction des ressources naturelles, pour la préservation des terres agricoles et, plus largement, pour le maintien des populations locales sur leurs lieux de vie,

? Admettons ensemble que les renoncements capacitaires des dernières décennies expliquent les fragilités structurelles que subissent aujourd'hui nos armées. C'est donc un soulagement pour nos armées que le Président de la République ait souhaité réparer ces fragilités, je remercie la ministre des armées, Florence Parly, qui a agi avec détermination pour que le cap soit tenu. Monsieur le Premier ministre, vous venez de rappeler les chiffres : ces trois dernières années, l'effort de défense a été conforme à la trajectoire budgétaire prévue par la LPM.

et de matériels : elle est avant tout une vision et une projection dans l'avenir de la place de la France dans le monde. C'est pourquoi cette LPM s'est attachée à répondre au mieux à un contexte géopolitique alarmant, dont la caractérisation dans la revue stratégique de 2017 a été confortée dans l'actualisation stratégique de 2021. Cela confirme la pertinence des priorités identifiées dès 2017 ainsi que des derniers ajustements destinés à prendre en compte l'actualité récente. Cette LPM s'inscrit dans le temps long. Elle garantit à la France les moyens d'une crédibilité qui soit à la hauteur de ce qu'elle est : une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est aussi pourquoi cette loi porte haut les couleurs de l'Europe, au service d'une autonomie stratégique européenne. Je pense par exemple à la dynamique créée par la responsabilisation accrue des Européens dans le cadre de l'Alliance atlantique. Dans une Union européenne à la recherche de sa boussole stratégique, la France a agi sans rechigner en faveur de l'Europe de la défense. D'ailleurs, notre commission des affaires étrangères n'a pas manqué de soutenir cette action, en appelant à un ambitieux fonds européen de la défense. Je regrette

pourtant la concrétisation d'une défense européenne que nous appelons de tous nos voeux. Elle renforcera utilement l'interopérabilité entre nos forces armées, car il n'est plus possible de continuer avec une telle fragmentation des systèmes d'armement entre Européens. Les préoccupantes provocations de la Turquie en Méditerranée orientale ont elles aussi guidé de tels choix. Y opposer un discours souverainiste trahit une faiblesse de vision stratégique à long terme. Vous-même, monsieur le président de la commission, avez déclaré : « Nous consentons très volontiers à cet effort », car il s'agit « d'un signal fort, mais aussi d'un acte fort, dont la portée opérationnelle doit être soulignée ». Avec cette programmation militaire, nous faisons le choix stratégique de l'innovation, du renseignement, de la cybersécurité, mais aussi du spatial, ce champ « assumé de rivalité stratégique permanente, voire de conflictualité

de soutien ; nous devons poursuivre l'effort de redressement et de modernisation de notre armée et maintenir un cap budgétaire ambitieux dans le grave contexte de récession économique que nous connaissons. Nos armées ont besoin que nous soutenions le choix fait par le Gouvernement d'une base industrielle et technologique de défense forte,

Cet effort est pleinement justifié et compris par la majorité d'entre nous au regard des turbulences géopolitiques pointées dans la revue stratégique de 2017 et toujours à l'oeuvre. Sur le plan comptable, où en sommes-nous aujourd'hui ? Si l'on s'en tient au budget de la défense que nous avons voté à la fin du mois de décembre dernier- c'était, pour moi, le premier -, il faut reconnaître que la trajectoire a été une nouvelle fois respectée, avec 39,2 milliards d'euros de crédits approuvés pour 2021.

-à préparer et à garantir un modèle d'armée complet à même d'intervenir sur tous les fronts, de la terre jusqu'à l'espace, au service de la sécurité de nos concitoyens et des intérêts de la France.

Les orateurs précédents l'ont rappelé : le Sénat attendait le projet de loi d'actualisation promis par l'article 7 de la loi de 2018. Tel n'est pas le choix qui a été fait ; c'est regrettable. Vous en avez exposé les raisons

Quant à la Russie, dont nous n'occultons pas la grande « stratégie byzantine » aux effets délétères, elle est un partenaire à bien des égards- je pense, par exemple, à la lutte contre le terrorisme -, ce qui nous invite au maintien d'un dialogue constant avec Moscou. Un équilibre doit être recherché. À l'issue du prochain Conseil européen, nous devrions en savoir un peu plus sur la manière dont Josep Borrell compte mettre en oeuvre avec la Russie son triptyque « riposter, contraindre, dialoguer ».

plus globalement, de la progression du fondamentalisme islamiste. La situation en Afghanistan est particulièrement inquiétante. Au Sahel, malgré des succès certains sur le terrain et l'engagement exemplaire des milliers de militaires français dans la bande sahélo-saharienne, la persistance d'États faillis complique la tâche ; on peut notamment le déplorer au Mali. Dans ces conditions, les groupes terroristes se régénèrent plus vite que les États ne s'organisent. On peut certes regretter l'extinction de Barkhane, mais les conditions ne semblent plus réunies pour obtenir des avancées probantes sans mettre en danger nos soldats, dont la présence en outre parfois mal comprise par les populations locales. Au reste- vous l'avez précisé, monsieur le Premier ministre -, il ne s'agit pas de renoncer : la France devrait rester fortement engagée à travers l'internationalisation de Barkhane. du RDSE, cette formule convient, car elle acte une responsabilité plus collective dans la région. Je pense en particulier à nos partenaires européens impliqués au sein de la force Takuba. Sa montée en puissance est une bonne chose, même si nous n'ignorons pas les difficultés inhérentes à sa mise en place. La France ne peut plus rester seule en première ligne sur des fronts qui concernent la sécurité de toute l'Europe Je n'oublie pas les autres défis qui se posent à notre défense. Ils sont nombreux : les cyberattaques de plus en plus fréquentes- les précédents orateurs les ont évoquées -, la criminalité organisée, le risque sanitaire identifié en 2017 et devenu réalité en 2020 avec la covid, l'instrumentalisation politique de la pression migratoire par la Turquie et, depuis peu, par le Maroc, etc. Nous sommes dans une sorte de « brouillard de guerre », pour reprendre les mots de Clausewitz, avec ses ennemis invisibles et hybrides. Le général Lecointre l'a plusieurs fois rappelé devant notre commission des affaires étrangères : « Il n'y a aucune raison de penser que cette instabilité cesse d'ici dix ou vingt ans. » Aussi, à l'évidence, la France doit-elle maintenir ses capacités opérationnelles.

L'effort porté sur les armes individuelles, avec les livraisons substantielles de fusils d'assaut HK 416 F, et sur la rénovation de l'équipement du combattant mérite d'être souligné. Cet effort garantit la crédibilité de l'axe central de la loi de programmation- une loi à

Au rang des inquiétudes, en revanche, je partage certaines des observations exposées par la commission des affaires étrangères. Ainsi, nous souhaitons quelques éclaircissements sur les programmes qui font l'objet d'ajustements budgétaires, dont le cumul représenterait 1 milliard d'euros,

À plus long terme, l'effort budgétaire sera-t-il suffisant pour couvrir les nouveaux champs de conflictualité que deviendront, faute d'être régulés, l'espace et les fonds marins ? Toutes ces préoccupations appellent, entre le Gouvernement et le Parlement, une confiance mutuelle que la loi d'actualisation était susceptible de consolider.

mais aussi les évolutions du contexte géostratégique et le bouleversement des priorités qu'impose la crise pandémique pour la sécurité humaine mondiale. Mais le débat

dit, vous réduisez une fois encore le rôle du Parlement dans l'élaboration de choix nationaux fondamentaux. Escamoter le Parlement sur des sujets d'une telle importance est grave, d'autant que le contrôle parlementaire sur notre stratégie de défense est déjà largement limité par les prérogatives exorbitantes du chef de l'État. Engagement des opérations militaires extérieures, autorisation des exportations d'armes, dissuasion nucléaire : les domaines réservés réduisent beaucoup le rôle du Parlement,

La loi de programmation militaire prévoit une dépense globale de 295 milliards d'euros sur toute la période. D'après le rapport de notre commission des affaires étrangères, 198 milliards d'euros ont été programmés Il resterait donc 95 milliards d'euros à engager sur les deux dernières années pour porter à 50 milliards d'euros, en 2025, le budget militaire de la France, déjà passé à quelque 39 milliards d'euros cette année. Alors qu'à peine la crise du covid ralentie votre gouvernement reprend le refrain de la « maîtrise des dépenses publiques » contre les dépenses sociales, expliquez-nous ce que vous allez sacrifier pour atteindre un tel niveau de dépenses militaires Vous l'expliquez d'autant moins que, selon notre commission, les surcoûts à prévoir atteignent déjà 8,6 milliards d'euros, ce qui aurait dû être une raison supplémentaire de débattre du périmètre d'actualisation. Il semble d'ailleurs que l'amélioration de la condition de nos militaires, les équipements « à hauteur d'homme » pour nos soldats et le maintien en condition opérationnelle, dont nous étions convenus de la nécessité lors de l'adoption du projet de loi de programmation, servent d'ores et déjà de variables d'ajustement.

même que la privatisation croissante de nos industries d'armement affaiblit le contrôle nécessaire de la Nation et fait s'envoler les coûts. Les enjeux d'une loi de programmation d'une telle ampleur ne peuvent être examinés en faisant abstraction des concepts stratégiques qu'elle entend servir. Depuis 2017, le discours présidentiel n'a cessé de renforcer l'affirmation selon laquelle notre sécurité ne saurait être assurée qu'avec un « modèle d'armée complet sur tout le spectre d'intervention davantage capable d'« entrer en premier » dans des conflits de « plus en plus haute intensité ». La montée des menaces justifierait donc une armée de plus en plus tournée vers la projection de nos forces. Or, au moment même où vous réaffirmez ce modèle de projection, l'échec de l'opération Barkhane au Sahel sonne comme un rappel à l'ordre. Nous y avons pourtant englouti progressivement plus de 1 milliard d'euros par an. Notre assemblée, qui a moult fois sollicité auditions et débats pour examiner et évaluer le bilan réel de cette intervention militaire d'envergure, a appris par la presse le revirement présidentiel sur Barkhane. Là encore, quel mépris du Parlement ! Pour notre part, nous n'avons cessé de donner l'alerte. Nous étions face à un engrenage : la militarisation risquait de créer un terrain propice à l'extension des menaces djihadistes, lesquelles prospèrent dans le chaos créé par la guerre dans des pays d'Afrique toujours pillés et vulnérables à la déstabilisation. Malheureusement, nous y sommes ; les violences s'étendent partout en Afrique- au Mali, au Burkina Faso, dans la région des trois frontières, en Côte d'Ivoire ou encore au Mozambique. Puisqu'il faut bien décrypter ce que l'on refuse de venir nous expliquer au Parlement,

ces milliards ne sont-ils pas indispensables à la sécurité du monde ? Notre priorité militaire peut-elle véritablement tenir lieu de politique de sécurité planétaire ? Ne faudrait-il pas au contraire travailler à de nouvelles logiques de développement et de coopération, qui fassent reculer le moins-disant fiscal qui confortent la mobilisation des ressources internes de ces pays ? Si nous ne nous donnons pas les moyens d'une lutte ambitieuse contre la pauvreté, la sous-alimentation, les dérèglements climatiques et toute forme d'insécurité humaine dans le monde, il y a fort à parier que la militarisation croissante de nos relations internationales n'engendrera ni paix, ni sécurité collective, ni recul des formes de guerre hybrides ou asymétriques. Bien au contraire, elle entraînera la dissémination des violences et des conflits. ne parle pas des ventes d'armes, dont nous sommes un champion mondial : elles dispersent un peu partout dans ce monde instable des arsenaux qui sont de véritables bombes à retardement, comme on l'a vu récemment au Yémen. Ainsi, tout nous incite à réinterroger les objectifs de la LPM. Nous prétendons créer de la sécurité mondiale en développant notre capacité militaire de projection dans tous les domaines. Nous le faisons en revendiquant le concept, élaboré par l'OTAN, des 2 % de dépenses militaires dans les budgets nationaux des pays de l'Alliance atlantique. Nous courons sur tous les fronts de l'escalade armée

en Afrique, comme je l'ai dit. Nous nous apprêtons à lancer le projet d'un porte-avions de nouvelle génération à propulsion nucléaire, estimé à 10 milliards d'euros d'ici à 2038, pour quels objectifs ? La sécurité de nos espaces maritimes ? Ou bien plutôt dans une logique de puissance et de projection, là encore, de nos forces extérieures ? Nous jouons un jeu dangereux en usant de notre puissance militaire comme d'une arme politique et diplomatique, loin de nos besoins de sécurité nationale.

pour la France, le Royaume-Uni ou l'Italie, l'urgence est toutefois d'adopter au plus vite de nouvelles mesures qui répondent aux préoccupations les plus aiguës. » En d'autres termes, on a préféré mettre le doigt et même les deux mains dans une machine dont on sait qu'elle nous happera le bras. Nous sommes les acteurs d'une escalade militaire mondiale qui est repartie à un rythme fou, tout autant tirée par les appétits de profits que font miroiter la sophistication et les ruptures technologiques

Ce cycle apparaît de nouveau sans fin. Loin du fatalisme de la guerre et des menaces, la France, tout en assurant sa sécurité, devrait lever haut et fort le drapeau de la désescalade. Or nous ne sommes jamais au rendez-vous des batailles mondiales pour le désarmement. Un vent de mobilisation s'est levé aux Nations unies pour relancer un processus mondial de désarmement militaire, avec la signature par de nombreux pays du traité sur l'interdiction des armes nucléaires nous avons combattu cette dynamique plutôt que de nourrir le débat mondial et multilatéral en faveur de nouvelles étapes de désarmement nucléaire. À son terme, la LPM aura consacré plus de 37 milliards d'euros à la modernisation de notre dissuasion. Or agir pour débarrasser le monde et notre pays de ce fardeau dans un processus multilatéral de désarmement reste une condition de la sécurité collective et de la paix. vous l'aurez compris : les élus de notre groupe s'opposeront au quitus que vous nous demandez, parce que de tels engagements budgétaires ne peuvent être ratifiés à la légère, encore moins aujourd'hui qu'hier, et parce que nous avons plus que jamais besoin de repenser les concepts mêmes de défense nationale et de sécurité humaine globale planétaire. On ne saurait les considérer, ces concepts, au seul prisme de la progression de nos dépenses militaires

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, mes chers collègues, en 2018, lors de l'examen initial de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025, le Sénat a unanimement salué l'effort sans précédent souhaité par le Gouvernement en matière de défense nationale. La LPM fixe de réelles ambitions pour nos forces, en tirant les enseignements d'un contexte stratégique marqué par l'augmentation et l'intensité des menaces. Après de nombreuses années de déflation et d'une réduction de moyens incohérente au regard de l'engagement de nos armées en opérations extérieures, cette loi de programmation a permis de réparer certaines fragilités et de préparer, à l'horizon de 2030, la défense de notre Nation et de l'Europe tout entière, grâce à une trajectoire de remontée en puissance. Les quatre axes prioritaires de la loi de programmation ont été validés et confortés par le Sénat : l'amélioration des conditions d'exercice de nos militaires, le renouvellement des capacités opérationnelles, le renforcement de notre autonomie stratégique dans les domaines de l'espace, du cyber et du renseignement, ainsi que le défi de l'innovation pour faire face aux enjeux à venir. À ces points de vigilance, le Sénat a souhaité ajouter une « clause de revoyure » afin de suivre, année après année, la trajectoire budgétaire et le calendrier des livraisons.

afin d'être prêts à remplir notre rôle lorsque le projet de loi d'actualisation nous serait soumis. Ainsi, dès la préparation du débat budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2021, nous avons engagé et multiplié les auditions. Nous nous sommes parfois sentis bien seuls à travailler sur ce sujet, sans nous défaire jamais de l'impression que des consignes de non-communication avaient été transmises. Comment expliquer autrement que des questions liées à la trajectoire de remontée de la préparation opérationnelle et à sa conformité aux objectifs fixés par la LPM n'aient pas obtenu de réponse ? Vous l'aurez compris, monsieur le Premier ministre, le Sénat n'est pas disposé à accepter que l'actualisation de la programmation militaire se réduise au seul débat que nous avons aujourd'hui.

nos soldats ne sont pas suffisamment entraînés par rapport aux standards internationaux et la remontée de l'activité opérationnelle a été reportée à 2025, alors que cette dernière est essentielle à leur sécurité en OPEX. Nous ne pouvons que constater que certains indicateurs ne progressent pas, même s'il est difficile d'apprécier si les moyens mis à la disposition de nos armées sont adaptés aux efforts à produire. Lors de nos déplacements, nous mesurons les attentes de nos marins, de nos aviateurs et de nos soldats, dont nous saluons l'engagement exceptionnel ; nous mesurons également leur satisfaction de voir arriver le premier sous-marin de classe Barracuda, les avions ravitailleurs A330 MRTT (), les premiers Griffon

la fixation d'objectifs annuels de progression de l'activité opérationnelle et la présentation d'un bilan annuel de remontée de la préparation opérationnelle. Aucune de ces deux dispositions n'a été mise en oeuvre. Notre travail préparatoire nous a permis d'estimer que les trajectoires de remontée de la préparation opérationnelle, non transmises, ne sont pas respectées. À titre d'exemple, les équipages des chars Leclerc ont vu la durée de leur entraînement diminuer de 35 % entre les deux premières années d'application de la loi de programmation. conditions, comment atteindre les objectifs de haute intensité à l'horizon de 2030 en prenant en compte l'actualisation stratégique ? Là encore, les discours qui tendraient à reporter à la prochaine LPM l'accélération de la préparation opérationnelle en vue de la haute intensité ne sont pas compatibles avec la réalité des faits. La haute intensité ne sera atteinte que si la trajectoire est mise en oeuvre suffisamment tôt, avec exigence et régularité. J'en arrive à l'entretien programmé des matériels (EPM), qui doit bénéficier de 35 milliards d'euros sur la durée de la LPM, dont 22 milliards d'euros

D'autres sont structurels et découlent de la mise en oeuvre de la politique de verticalisation des contrats d'entretien programmé des matériels, notamment dans le domaine aéronautique. Ces contrats verticalisés se traduisent dans un premier temps par des surcoûts en raison de la création de nouvelles chaînes industrielles d'EPM et de la remise à niveau des stocks de pièces de rechange étatiques, transférés à l'industriel lors de la mise en oeuvre du contrat verticalisé. Ainsi,

la dotation budgétaire dédiée à l'EPM devant atteindre 6,5 milliards d'euros. De tous ces sujets, monsieur le Premier ministre, nous aurions pu et dû débattre longuement, sans oublier les services de soutien de nos armées, essentiels, dévoués, cultivant l'excellence malgré des conditions difficilement tenables. Comment peut-on voir se creuser encore, en pleine pandémie, le déficit en médecins de premier recours ? Comment peut-on atteindre des taux de projection des équipes chirurgicales supérieurs à 200 % ? % ? Vous le voyez, les sujets ne manquent pas ; ils sont d'une importance cruciale pour nos forces, ce qui justifie pleinement notre exigence d'un débat parlementaire approfondi. Les efforts engagés par le Gouvernement pour nos armées sont reconnus par le Sénat. Il serait souhaitable que le Gouvernement reconnaisse réciproquement le rôle du Parlement sur ces sujets. Tout à fait ! Certes, la défense est vue comme un domaine régalien, mais le lien entre la Nation et son armée est plus important que jamais, alors que la pandémie a mis notre pays dans une situation économique préoccupante. Pour conclure, je souhaite évoquer la réduction du format de l'opération Barkhane. Autre sujet, même méthode : c'est par la presse et les réseaux sociaux que nous avons appris, le 10 juin dernier, la volonté du Président de la République, après un deuxième coup d'État au Mali, de redimensionner et de revoir les modalités d'engagement de nos forces au sein de Barkhane

Chacune de ces morts est une plaie ouverte pour nous tous, car, même si nous n'avons eu à nous exprimer qu'une seule fois, par un vote sur l'envoi de nos soldats français au Mali, nous avons bien donné l'autorisation requise par l'article 35 de notre Constitution à cette OPEX.

Ne nous y trompons pas, nous n'avons qu'un seul objectif : donner à nos forces armées les moyens de faire face à leurs engagements.

cela a été dit et répété : le Sénat avait adopté la loi de programmation militaire 2019-2025 à une très large majorité des groupes politiques,

pourquoi ne pas procéder à une actualisation législative de la loi de programmation militaire ? Est-ce par crainte de vous confronter au Parlement ou est-ce simplement pour nous signifier votre mépris que vous avez choisi de sacrifier à la pire tradition des pratiques autoritaires et antiparlementaires de la V République ? Je vous le dis : cette décision de contourner le Parlement déshonore et discrédite le Gouvernement, et ce pour plusieurs raisons. Cette décision est tout d'abord une erreur de droit. En effet, l'article 7 de la LPM prévoit explicitement une actualisation en 2021. Je vais me permettre, monsieur le Premier ministre, de vous en donner lecture, au cas où vous ne l'auriez pas bien lu : « La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en oeuvre avant la fin de l'année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière

Un débat n'a pas force de loi ; vous faites donc le choix, dans un État de droit, de vous asseoir sur un texte pourtant adopté à une très large majorité par le Parlement. Si cette décision est une erreur de droit, elle est aussi une faute politique.

davantage de consultation du Parlement, alors que ce dernier doit approuver tout engagement extérieur de plus de quatre mois, justifie à lui seul la nécessité d'un débat sur la LPM. C'est une faute politique que de refuser de consulter le Parlement sur une politique publique aussi majeure et stratégique que la défense de la Nation.

fait défaut à la ministre des armées. Nous avons adopté très largement la LPM et nous avons voté, dans les projets de loi de finances successifs,

pour la période 2019-2023. Le même article prévoit en outre que les « crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d'arbitrages complémentaires

Autrement dit, les exercices 2024 et 2025 ne sont pas couverts par cette LPM. Ainsi, en programmation, ce sont environ 97 milliards d'euros qui passent à la trappe,

de la LPM reporte l'essentiel de l'effort à la fin de la période, l'annulation de l'actualisation rend très hypothétiques les quelque 4 500 créations d'emplois prévues entre 2023 et 2025. Je souhaite enfin apporter quelques précisions sur vos renoncements par rapport aux objectifs fixés, dans la mesure où le Gouvernement raisonne à enveloppe budgétaire constante.

deux risques majeurs pesant sur la trajectoire financière : les OPEX et l'export d'armement. Le désengagement de Barkhane est un processus qui ne peut être que progressif, tant sur le plan opérationnel que sur le plan budgétaire.

le soutien aux exportations, deux difficultés se font jour : d'une part, la cession de matériels d'occasion, prélevés sur le parc existant ; d'autre part, l'accélération de certaines commandes de matériel neuf à soutenir le plan de charge des entreprises de notre base industrielle et technologique de défense. Si cet effort contribue à la pérennité et à l'autonomie stratégique de notre industrie de défense,

J'en arrive aux renoncements qu'implique cette actualisation. L'absence d'une véritable transparence sur les arbitrages défavorables nous oblige à

Il est regrettable que l'exigence de transparence envers le Parlement sur l'ensemble de ces points ne soit pas respectée. Le contrôle parlementaire est indispensable au succès de l'action militaire du Gouvernement. Nous regrettons sincèrement que votre gouvernement

nous étions prêts à agir autrement -, de voter contre votre déclaration. Je souhaite que mes derniers mots soient pour nos soldats. Puissent-ils entendre l'hommage que le Sénat leur rend, et qu'ils soient assurés du soutien et de l'engagement sans faille des sénateurs socialistes à leurs côtés. La parole

Nous vous avons bien écouté, monsieur le Premier ministre, mais nous n'avons été ni convaincus ni rassurés. Nous attendions le dépôt, en 2021, d'un véritable projet de loi, assorti d'une étude d'impact et tirant les enseignements de l'actualisation de la revue stratégique. Au lieu de cela, que nous proposez-vous ? Pour préparer ce débat, vous avez transmis aux groupes politiques un document intitulé, qui s'apparente davantage à une plaquette de communication qu'à une présentation chiffrée et exhaustive des choix et ajustements opérés par la ministre des armées. Cette méthode est pire que tout Vous nous demandez de nous prononcer sur le bilan de votre action depuis 2019 et de soutenir- je cite la note d'accompagnement -« la poursuite de la remontée en puissance de nos forces armées ».

car réduire le débat sur l'actualisation à un soutien ou non au Gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Le président Cambon l'a rappelé : le Sénat a massivement approuvé les objectifs de la loi de programmation militaire à l'horizon de 2025 et, au-delà, vers l'Ambition opérationnelle 2030.

à une appropriation et à une approbation par le plus grand nombre ? C'est la définition même de la démocratie représentative ... À laisser le débat se tenir dans un cercle fermé, les sujets de défense deviennent suspects. À étouffer le débat et à le réduire à un exercice de communication sans pédagogie ni contradiction, la défense pourrait se résumer, dans l'esprit des non-initiés, à un boulet budgétaire pour la Nation. Cette absence de dialogue conduit la société civile à remettre en cause les choix et les orientations de notre pays. Or, à l'heure où la menace est protéiforme et où l'affrontement se produit dans de multiples domaines, nous voilà bloqués dans une impasse, la faute à un État gestionnaire et technocrate plus que visionnaire et stratège. Ce constat est d'autant plus surprenant et décevant que l'évolution du contexte sécuritaire justifie un effort plus grand de la Nation. Pourtant, le champ des possibles et les marges de manoeuvre de nos armées sont très réduits. Vous l'aurez compris, je m'associe pleinement aux conclusions exposées par le président Cambon quant à l'absence de transparence du Gouvernement et à l'ampleur des ajustements mis en oeuvre par la ministre des armées. Ce que nous avons fait sous la forme d'un rapport d'information, avec les moyens du bord- tous les intervenants avant moi l'ont rappelé -et en procédant par déduction à partir des réponses parcellaires et parfois volontairement lacunaires de nos interlocuteurs, aurait mérité de prendre la forme d'un rapport législatif. Si cette LPM devait être « à hauteur d'homme », elle devait surtout être à la hauteur de la menace qui sourd et de l'histoire qui s'écrit dans la bande sahélo-saharienne, en Méditerranée orientale, dans le Haut-Karabagh, en Libye ou sur les frontières plus immatérielles de l'innovation et des technologies duales telles que les drones-

des reports, voire des renoncements, sur certains objectifs fixés pour 2025. Je fais référence aux bâtiments de guerre contre les mines,

ce que la loi fait, seule la loi peut le défaire, sauf à nier ce qui fait le coeur de notre démocratie parlementaire ! Ensuite, c'est par un travail de déduction, qui n'est pas digne de la relation de confiance qui doit s'établir entre le Parlement et l'exécutif sur des sujets d'une telle gravité, que nous nous sommes rendu compte que le périmètre des ajustements budgétaires dépassait très largement le milliard d'euros annoncé par le Gouvernement. En réalité, les ajustements annuels opérés de 2019 à 2021 représentent déjà 3,1 milliards d'euros, qui sont fléchés vers des programmes à effet majeur jugés- à juste titre -prioritaires : le renseignement, la détection et les services spatiaux, le numérique et la cyberdéfense, la rénovation et la prolongation de la durée de vie des chars Leclerc et le lancement des études de propulsion nucléaire du futur porte-avions de nouvelle génération, qui doit entrer en service en 2038. Je n'oublie pas non plus l'effort budgétaire supplémentaire réalisé en faveur du volet hébergement du plan Famille. Là encore, nous sommes loin du compte, puisqu'il faut ajouter à ces ajustements le surcoût des OPEX- 600 millions d'euros rien que pour 2019 et 2020 le reste à charge de la cession des Rafale à la Grèce et à la Croatie, sur lequel aucune donnée ne nous a été communiquée, l'achat d'une frégate de défense et d'intervention (FDI) supplémentaire et des dépenses de soutien et d'imprévus telle la réparation du SNA, qui, soit dit en passant, est une prouesse à saluer. Au total, sur le fondement d'estimations prudentes, nous constatons que ces ajustements représentent près de 7,4 milliards d'euros. Si l'on y ajoute le coût prévisionnel de l'entretien programmé des matériels, le respect de la trajectoire de remontée de la préparation opérationnelle à l'horizon de 2025 et les moyens qui devront être déployés pour atteindre la haute intensité en 2030, c'est sur un périmètre minimal de 8,6 milliards d'euros qu'aurait dû porter l'actualisation. Soyons clairs, il s'agit d'un simple constat. Ce que nous dénonçons, ce ne sont pas ces ajustements, qui peuvent tout à fait être justifiés ; c'est le manque de transparence sur les concessions qui devront être faites par ailleurs pour financer ces efforts. À l'heure du « quoi qu'il en coûte », devenu un mantra plus dangereux qu'utile pour notre pays lourdement endetté, comment comprendre que, dans un domaine de l'action publique où l'effort est indispensable car imposé par la réalité du monde, votre gouvernement rogne les dépenses militaires, qui plus est en catimini ? Notre méthode de travail, celle qui consiste à analyser le fond avant de prendre position, démontre bien que le Gouvernement doit travailler avec le Parlement, de manière sincère et transparente.

la réduction capacitaire ne trouve pas de réponse à ce stade, comme le chef d'état-major des armées- je veux moi aussi lui rendre hommage -nous l'a confirmé en commission, sauf à améliorer l'activité du parc existant et à prolonger, le cas échant, la durée de vie des Mirage 2000-5, au prix d'un surcoût en EPM et en Quant à la dimension financière de l'opération, il s'agit de céder des appareils opérationnels qu'il faudra remplacer au prix du neuf ; le modèle économique de ces partenariats stratégiques atteint donc déjà ses limites Par ailleurs, bien qu'il faille se féliciter du nouveau succès à l'export du Rafale en Indonésie, en version neuve cette fois, ce n'est pas un problème de coût qui se posera à l'armée de l'air, mais bien celui du calendrier de livraison des futurs avions par Dassault, qui ne dispose que d'une seule chaîne de montage de Rafale- je rappelle qu'il faut trois ans entre une commande et une livraison. Je regrette en outre que l'ambition d'une LPM « à hauteur d'homme » soit remise en cause par les retards de livraison sur les véhicules blindés légers et les véhicules des forces spéciales. Ces programmes s'avèrent déterminants pour la sécurité et la protection de nos soldats en OPEX, comme vous l'avez fort justement rappelé, monsieur le Premier ministre. Les véhicules blindés légers, du fait des missions de reconnaissance et de liaison sont particulièrement exposés aux risques balistiques, aux mines et autres engins explosifs improvisés (EEI). Or le retard pris dans la régénération des VBL semble acté dans l'actualisation de 2021.

La même question peut se poser pour le véhicule qui remplacera l'engin blindé du génie en matière de lutte contre les risques de mines et autres EEI. Il y va de la protection individuelle de nos militaires. On ne saurait se satisfaire que de tels retards soient imputés à des problèmes industriels. D'ici à 2025, il reste quatre ans pour exiger que le retard soit rattrapé ; monsieur le Premier ministre, il s'agit d'une demande que je vous adresse solennellement aujourd'hui, permettez-moi de vous livrer le fond de ma pensée. Le Gouvernement a raté la dernière occasion qui lui était offerte avant 2022 de présenter dans de bonnes conditions les efforts d'adaptation de nos armées à l'environnement international plus menaçant et imprévisible qui nous entoure. Nous ne voudrions pas que cette loi de programmation militaire souffre des mêmes syndromes que les grandes réformes portées par votre gouvernement, à savoir le syndrome de la déconnexion entre les déclarations et les actes et les ravages de la politique du « en même temps ». En début de LPM, le Président de la République annonçait que la dissuasion était sanctuarisée, que le développement des capacités dans le domaine du cyber était une priorité, tout comme le renseignement, et j'en passe. Or, quand tout devient prioritaire, plus rien ne l'est. ne l'est. Et les priorités politiques ont fini par prendre le pas sur les priorités opérationnelles. Les programmes à effet majeur sont devenus des objets politiques avant d'être des réponses à des besoins opérationnels. Cette mainmise du politique sur les affaires militaires a stérilisé l'échelon interarmées et réduit les états-majors au rôle de sténographes de la pensée complexe. L'État stratège n'est pas celui qui réactualise en catimini pour pouvoir revenir sur la parole donnée l'État stratège n'ambitionne pas de réorienter ce qu'il ne pourra pas respecter. L'État stratège est celui qui voit loin, qui associe, qui croise et qui capitalise. capitalise. Il milite pour un échelon interarmées maître de son destin, ayant les moyens d'anticiper, de se préparer et de se réformer pour faire face aux ruptures actuelles et futures. C'est pourquoi, s'il y a des dépenses supplémentaires, il faut discuter de manière lucide et en toute transparence des économies ou des sacrifices à réaliser par ailleurs. Nous le devons aux militaires, femmes et hommes qui, pour notre sécurité, mettent leur vie en danger. Ils méritent notre indéfectible soutien.

passion pour la vie parlementaire et pour le contrôle que nous exerçons. Pourtant, cette passion n'a absolument rien à voir avec l'importance que j'accorde, monsieur le Premier ministre, aux relations multiséculaires entre la France et son armée. Je ne suis pas un gaulliste historique, cher Roger, ... Regrets

au vélo-cargo et aux pistes cyclables en milieu périurbain qu'aux 295 milliards d'euros de la loi de programmation militaire.

pour évaluer toutes les variations des caractères, combien le président de la commission des affaires étrangères et de la défense nationale, ainsi que tous les membres de cette commission, étaient choqués

Je ne reviendrai pas non plus sur l'intervention brillante de mon jeune collègue Cédric Perrin, qui maîtrise absolument ces dossiers. Je voudrais simplement vous saisir, monsieur le Premier ministre,

Madame la ministre, vous ne l'aviez sans doute pas pressentie, puisque nous ne l'avions pas évoquée durant ce débat auquel vous avez participé. Vous aviez donc l'occasion, au travers d'un débat parlementaire, de rétablir le lien de confiance et de compréhension entre un Parlement, en tout cas un Sénat, qui soutient pour l'essentiel cette action, et votre action elle-même, qui doit s'adapter à l'environnement. Permettez-moi de prendre pour exemple la « mort cérébrale » de l'OTAN. Il se trouve que l'OTAN a choisi- j'y vois une victoire diplomatique pour la France -de se réunir à Paris pour annoncer son nouveau programme. Dans un communiqué interminable, tout

la Turquie, membre de l'OTAN, qui compromet notre vision collective européenne en Syrie, en Méditerranée orientale ainsi qu'au Caucase, naturellement, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

la politique de l'OTAN consistant à faire de la Russie l'ennemi que vous aimerez haïr ? Je pense profondément qu'un débat parlementaire aurait permis d'approfondir ce sujet et que des leçons

du superficiel, de l'émotif, du spectaculaire et du tirage au sort. Je préfère l'élection et, d'ailleurs, les électeurs nous préfèrent- nous venons de le voir. Je n'ai pris que sept minutes, parce que je n'avais que cela à dire, l'essentiel ayant été exprimé avec compétence par des collègues qui ont la passion de ces sujets.

des surcoûts liés aux opérations extérieures. Cela me donne l'occasion de m'associer à l'hommage rendu à nos soldats par de nombreux orateurs avant moi. Chaque année, nous votons une dotation budgétaire destinée à couvrir

se rapproche des besoins grâce à l'augmentation progressive de la dotation initiale : de 850 millions d'euros, elle est passée à 1,1 milliard d'euros, Les besoins de financement additionnels, c'est-à-dire les surcoûts nets non couverts par la dotation initiale, ont essentiellement été financés par un recours à la réserve de précaution. cet égard à saluer l'effort de transparence et de sincérité budgétaire accompli par le ministère des armées. Dans son rapport sur le budget de l'État en 2020, la Cour des comptes considère que l'aboutissement de la trajectoire de la dotation a mis un terme aux sous-budgétisations chroniques des surcoûts OPEX. L'intégration des dépenses liées aux missions intérieures au sein de la dotation initiale a également contribué à l'amélioration de la programmation de ces coûts. Afin de parachever ce mouvement, la Cour des comptes recommande d'inclure dans la dotation initiale les dépenses de personnel liées aux opérations intérieures telles que l'opération Sentinelle.

Malgré l'amélioration de la programmation budgétaire des surcoûts, la majorité sénatoriale reproche au Gouvernement de ne pas recourir à la solidarité interministérielle pour couvrir ces surcoûts nets. Cette critique ne me semble pas justifiée, dans la mesure où les crédits de la réserve de précaution sont interministériels. De surcroît, au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles nous faisons face, il paraît difficile de faire jouer cette solidarité interministérielle au-delà de la mobilisation de la réserve de précaution. Que dirait-on si l'on prélevait des crédits destinés à la santé, à la vaccination ou à l'action sociale pour financer ces OPEX ? Force est de constater que les efforts déployés par le Gouvernement tranchent nettement avec l'inaction des gouvernements Raffarin, Villepin et Fillon. Ces gouvernements n'ont, en effet, rien fait pour mettre fin à la sous-dotation des surcoûts OPEX. Voilà un discours les besoins de financement additionnels par des annulations de crédits d'équipement des forces, alors même que la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 disposait que ces surcoûts devaient être financés par la réserve de précaution interministérielle. Au total, près d'un milliard d'euros d'équipement des forces ont ainsi disparu. À l'époque, j'ai entendu peu de litanies sur la chute de notre dotation à l'armée La majorité sénatoriale est d'autant plus mal placée pour donner des leçons que le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été marqué par une baisse des budgets annuels de 2 milliards d'euros entre 2009 et 2012, par la fermeture de quatre-vingt-trois emprises militaires et par la suppression de près de 60 000 emplois militaires. Eh oui ! Avant de conclure, je souhaite saluer la décision du Président de la République relative à la reconfiguration de l'opération Barkhane. Cette décision est bienvenue : elle participe d'une logique d'européanisation et d'internationalisation de la lutte contre le terrorisme, en somme de meilleur partage du fardeau. À cet égard, je souhaite savoir comment la transformation je souhaite savoir comment la transformation du dispositif militaire français au Sahel se traduira sur le plan budgétaire. Pour ces raisons, monsieur le Premier ministre, notre groupe soutiendra votre déclaration. La parole

et de dialogue permanent avec la ministre, qui prévaut jusqu'à ce jour. Entendez, dès lors, notre incompréhension totale, exprimée par notre collègue Gérard Longuet, face au choix assumé que vous faites de ne pas respecter l'article 7 de la loi que nous avons adoptée, tout en rappelant, par ailleurs, que vous respectez le Parlement.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir prévu un vote sur un projet de loi d'actualisation plutôt qu'un blanc-seing politique ? Nos militaires, comme nos industriels, d'ailleurs, n'attendent pas des indications, mais des engagements chiffrés ; surtout, ils attendent de savoir que ceux-ci seront respectés, comme ce fut le cas depuis trois ans. Nous nous réjouissons de la bonne exécution de la LPM, mais l'actualisation nous aurait offert des garanties concernant l'exécution à venir. L'incertitude de la courbe du PIB, que vous avancez comme argument, devrait au contraire nous convaincre de sécuriser la trajectoire budgétaire de la défense pour les années 2024 et 2025. Ce débat est un rendez-vous raté. Notre soutien était acquis à une véritable discussion sur les ajustements à apporter en cours de programmation. Nous souhaitions accompagner des décisions parfois difficiles, parce que nous les comprenons, et continuer tout simplement à travailler dans la confiance et la transparence sur les enjeux majeurs que sont l'amélioration opérationnelle, la disponibilité des équipements, l'évolution des effectifs et le respect de la trajectoire financière. est du bilan, au tiers du parcours de la LPM, les réponses partielles du ministère des armées nous ont confirmé ce que nous savions déjà, à savoir qu'il existe des besoins nouveaux et que ceux-ci devront être financés à enveloppe constante. Certains grands projets financièrement très lourds seront probablement sanctuarisés : le renouvellement de la dissuasion nucléaire, le porte-avions de nouvelle génération ainsi que- nous le savons depuis quelques heures Mais nous craignons des effets d'éviction sur d'autres programmes, d'autant que l'apparition de nouvelles menaces génère des besoins capacitaires dans les domaines spatial et cyber ou dans celui de la lutte anti-drones. Concernant l'armée de terre, le traitement des obsolescences du char Leclerc sera coûteux ; si l'on veut être prêt pour la haute intensité et réaliser l'Ambition 2030, cette remise à niveau devra se faire sans effet d'éviction sur d'autres aspects du programme Scorpion. Certes, les évolutions de la programmation sont naturelles dans un contexte stratégique fluctuant, s'agissant de programmes industriels lourds et technologiquement complexes. Mais nous avons besoin de clarté, monsieur le Premier ministre, sur les programmes sanctuarisés et sur ceux pour lesquels vous envisagez un ralentissement.

Il s'agit certes d'estimations, mais elles n'ont rien de fantaisiste : nous nous contentons de recenser des ajustements qui sont indiscutables. Si le Gouvernement n'est pas d'accord sur les chiffres, il lui appartient de mieux en informer le Parlement. également mettre l'accent sur l'un des objectifs majeurs de la loi de programmation : celui qui consiste à prendre en compte les besoins « à hauteur d'homme et de femme ». Les programmes à effet majeur sont indissociables des autres opérations d'armement qui visent à renforcer les équipements et la protection individuelle de nos soldats. Qu'il s'agisse de l'armement léger, de la vision nocturne ou des dispositifs de lutte contre les engins explosifs, l'effort d'équipement promis au titre de la LPM ne doit pas être relâché. Concrètement, un suivi tout particulier doit être accordé aux petits équipements, qui occupent une grande place dans la sécurité du combattant et doivent être préservés

Face à la menace des mines et des engins explosifs, nous demandons l'accélération de la livraison des kits de blindage commandés en urgence, afin de renforcer la protection des véhicules blindés légers. Comme l'a dit mon collègue Cédric Perrin, il faudrait aussi songer à ériger en priorité nouvelle le projet de véhicule blindé d'aide à l'engagement, ou VBAE, pour commencer à remplacer le VBL avant la fin de la LPM. Nous constatons des retards dans les livraisons du programme Scorpion. Nous pouvons également nous interroger sur notre autonomie en matière d'approvisionnement en munitions. Notre rapport d'information a mis en évidence la nécessité de chiffrer dès à présent les besoins en matériels et en préparation opérationnelle afin de remplir les objectifs de l'actualisation stratégique et de l'Ambition de l'Ambition 2030- ces besoins se chiffrent en milliards d'euros. La question des effectifs, c'est-à-dire de la fidélisation et de l'amélioration de la vie militaire, n'est pas accessoire par rapport à celle des équipements. Il y va au contraire de la valeur cardinale de nos armées, celle sur laquelle doit reposer le lien de confiance entre la Nation et ses forces armées- armées- nous en sommes tous ici convaincus, je le sais. C'est pourquoi il est dommage que nous ne puissions offrir en retour aux femmes et aux hommes qui nous protègent, et qui méritent mieux qu'une simple déclaration politique ou générale, une loi d'actualisation sécurisant leurs moyens et leur condition militaire. À cet égard, au nom de mon groupe politique, je m'associe pleinement à l'appel lancé en faveur du service de santé des armées. Il est urgent de doter ce service des personnels suffisants et d'offrir à nos médecins et infirmiers de meilleures conditions de vie, à la hauteur de leur engagement pour la Nation. Pour toutes ces raisons, qui s'ajoutent à celles qui ont déjà été évoquées par mon collègue Gilbert Roger, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat votera contre la déclaration du Gouvernement. La parole

on ne peut pas en même temps dire qu'on respecte le Parlement et se flatter de recourir systématiquement à l'article 50-1 de la Constitution, comme si le Parlement était une chambre d'enregistrement,

bouleverse les conditions de l'actualisation de la LPM, ce qui est reconnaître un bouleversement, et ne pas appliquer l'article 3, qui a justement été écrit pour que soit prise en compte l'évolution de la situation macroéconomique. On ne peut pas en même temps dire qu'on respecte la LPM et refuser d'appliquer deux de ses articles. On ne peut pas en même temps faire valoir le « quoi qu'il en coûte » pour répondre à la crise sanitaire et ne pas en tirer les conséquences pour nos forces armées. Monsieur le Premier ministre, madame la ministre, nul n'est au-dessus des lois, fût-il Jupiter. Ce n'est pas parce que le Gouvernement estime de façon unilatérale qu'il n'y a pas lieu de légiférer que le Parlement, souverain en la matière, doit se ranger sans discussion à cette appréciation. Il n'y a pas de place pour le « en même temps » quand il s'agit de la souveraineté de la France, de nos armées et de nos soldats qui sont exposés ; il n'y a pas de place pour le « en même temps » quand il y va des prérogatives de souveraineté nationale. Vous nous demandez de renoncer à une loi d'actualisation. Je ne peux imaginer un seul instant que vous ayez pu penser que nous étions disposés à troquer, pour solde de tout compte, un texte de loi qui nous engagerait, vous comme nous, contre un débat qui vous dédouanerait de vos responsabilités et réduirait le travail du Parlement à une simple forme d'enregistrement.

La LPM est l'outil indispensable au soutien de l'engagement politique du Président de la République en matière de défense : un plan de frappe de près de 300 milliards d'euros pour réparer et préparer nos armées. La loi de programmation militaire, c'est la réponse à une ambition, celle que le Président de la République a définie pour répondre aux enjeux d'un contexte stratégique- certains d'entre vous en ont rappelé les contours -marqué par une accentuation des tensions internationales, par la persistance de la menace terroriste et par l'affirmation désinhibée

Et comment en aurait-il été autrement ? Pendant des années, le budget des armées n'avait cessé de diminuer alors que, dans le même temps, les engagements de la France allaient croissant. Pendant des années, la défense avait été la variable d'ajustement des finances publiques. Voilà maintenant quatre ans que ce n'est plus le cas, et je m'en félicite. L'engagement de nos soldats, aviateurs et marins est constant et sans réserve. Nous devons donc être à la hauteur.

supplémentaires dans notre économie. Autrement dit, en quatre ans, nous avons apporté l'équivalent de deux années de budget d'investissement supplémentaires.

il y a les lois de finances initiales, mais il y a surtout l'exécution de ces lois de finances. Or, pour la première fois depuis des décennies, la LPM est respectée

à l'Assemblée nationale, au titre de l'année 2020, dans le cadre du « printemps de l'évaluation ». Et je ne doute pas, monsieur le président Cambon, que j'aurai encore à en rendre compte- c'est mon devoir - devant votre commission. Vous êtes

une formule que les anglophones affectionnent, la LPM « délivre ». Je ne détaillerai pas devant vous la longue liste des matériels qui ont d'ores et déjà été livrés à nos forces. Les matériels arrivent dans les unités ! Et nous constatons- vous constatez -chaque jour l'impact positif de ce changement sur le moral de nos militaires.

davantage : la guerre se gagne certes avec des matériels, mais elle se gagne surtout avec des femmes et des hommes servant notre pays avec courage et avec abnégation. précisément, la LPM 2019-2025 se caractérise par sa hauteur d'homme. Quand on attend de nos forces qu'elles s'engagent pleinement dans les missions qu'on leur a fixées,

près de 50 000 nouveaux fusils d'assaut ont été distribués, soit plus de 60 % de la cible ; 100 % des personnels déployés en opérations extérieures sont équipés du nouveau treillis ignifugé, plus protecteur que le précédent les nouveaux gilets pare-balles ont tous été livrés aux personnels qui devaient en être équipés. Certains d'entre vous ont mentionné- je les en remercie -le plan Famille il est extrêmement complet. Il a été mis en place pour faire face aux difficultés que rencontraient les militaires et leurs familles dans leur vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Les mesures retenues couvrent la condition du personnel, l'action sociale, la formation professionnelle, l'emploi des conjoints, le logement, l'hébergement Vous l'avez compris, le cap est tenu en direction d'objectifs que nous avions fixés ensemble en 2018. dois donc avouer ma perplexité à entendre ceux qui en leur temps avaient voté des coupes budgétaires massives

Qu'il faudrait une diminution du budget de la défense pour que leur vote soit favorable ? Que la hausse des moyens

! Je sais bien, cela vous gêne ! Allez-vous voter contre une meilleure protection des Français aujourd'hui et demain ? Contre le renouvellement des blindés, des frégates et des avions vieillissants de nos armées ?

d'atteindre 2 % du PIB à l'horizon 2025 pour nos armées. Or, si les ressources financières ont été fixées pour la première partie de la loi de programmation militaire, jusqu'en 2023 inclus,

Recourir à un texte législatif, mesdames, messieurs les sénateurs, eût été inopérant, car nous ne disposons pas de prévisions macroéconomiques fiables pour les années 2024 et 2025.

les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), la santé et la lutte anti-drones. Troisième axe : « mieux se préparer », concerne l'entraînement et la préparation opérationnelle. Les conflits d'aujourd'hui montrent que nos armées doivent être prêtes à riposter dans tous les champs de la conflictualité, qu'ils soient matériels ou immatériels, ce qui suppose un entraînement plus conséquent et plus sophistiqué ; l'effort en cours sur la disponibilité des matériels y contribue directement. Nous sommes donc bien en marche vers l'actualisation : nous travaillons à ce qu'elle puisse intervenir en temps utile.

ces montants ne représentent en aucun cas un surcoût net sur l'enveloppe de la LPM ». Nous voilà rassurés ! Je vais vous le dire, quant à moi, de manière plus claire : il n'y a pas de surcoût de 8,6 milliards

les rapports d'exécution que nous produisons chaque semestre à votre attention. Il semble que ce rapport de votre commission fasse référence à certains décalages.

il n'y a là aucun surcoût ! Nous avons simplement décidé d'anticiper d'une année la commande de la troisième frégate, qui était prévue avant la fin de la loi de programmation militaire. Où est donc le surcoût ? Il s'agit d'une décision qui permet d'assurer la continuité du plan de charge de Naval Group, à Lorient. En ce qui concerne les dépenses liées au covid, je me félicite de l'agilité dont le ministère des armées a su faire preuve en se mobilisant pleinement pour que tous les crédits qui ne pouvaient être dépensés en raison des retards de certains travaux puissent être redéployés. Nous avons donc accéléré la dépense partout où cela était possible, non pour le plaisir de dépenser l'argent public, mais bien pour répondre aux besoins de nos armées et pour soutenir notre économie au moment où elle en avait le plus besoin, en y injectant 1 milliard d'euros

historiques à l'exportation concernant le Rafale, je trouve extraordinaire qu'une excellente nouvelle pour nos emplois, pour nos entreprises et pour notre influence à l'international soit considérée par certains comme un problème. Pour ce qui est de l'export de Rafale à la Grèce, vous savez que cette commande se traduira par la production par Dassault de dix-huit avions neufs.

des appareils d'occasion : nous avons déjà passé la commande qui permettra de compenser l'impact de la cession d'appareils d'occasion aux armées grecques pour notre armée de l'air et de l'espace.

Là encore, contrairement à ce que j'ai pu entendre, et je m'en suis personnellement entretenue avec M. le président de la commission, ces appareils seront évidemment compensés à l'armée de l'air et de l'espace.

Entre 2009 et 2013, ce ne sont pas moins de 3,8 milliards d'euros qui ont manqué à l'appel si l'on compare les budgets exécutés à ce que prévoyait une LPM pourtant calculée au plus juste. Entre 2008 et 2015, 60 000 emplois ont été supprimés au sein du ministère de la défense. Ces suppressions ont pesé sur toutes les armées et sur tous les services de soutien

capacité, mais aussi à renouveler des équipements anciens dont le maintien en condition opérationnelle aurait été extrêmement coûteux.

mais que le coût du programme, lui, n'a pas varié ? Autrement dit, la marine nationale a acquis ces bateaux à un coût unitaire multiplié par deux.

qui en permettent l'exécution. Alors, ressaisissez-vous. Ça suffit ! Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'avez compris, la LPM est un engagement pleinement respecté par le Gouvernement. Nous ne dévions pas de la cible ; le cap est fermement tenu. Cette loi de programmation militaire, vous le savez mieux que quiconque, est une première étape vers l'Ambition 2030, vers le modèle d'armée complet, durable et équilibré qui permettra de protéger la France et les Français des menaces futures. Cet effort de remontée en puissance de nos armées, nous le poursuivrons bien évidemment au cours de l'année 2021 et à travers le budget pour 2022. Il est essentiel que la représentation nationale y apporte son plein soutien,

ce que vous faites ! À la demande du Gouvernement, le Sénat est appelé à se prononcer par un vote sur cette déclaration. Conformément à l'article 39, alinéa 6, de notre règlement, il va donc être procédé à un scrutin public ordinaire dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement ; aucune explication de vote n'est admise.

scrutin est clos.